les réserves d'usage. En application de l'article 28 de la Constitution, la session ordinaire de 2021-2022 est ouverte.

Le mandat de nos collègues a débuté vendredi 1 octobre, à zéro heure. Nous les accueillons au Sénat avec plaisir et leur souhaitons un excellent mandat. Acte est donné de cette communication. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, c'est une profonde tristesse qui nous a envahis quand nous avons appris, le 5 juillet dernier, la disparition de notre collègue Patrick Boré, sénateur des Bouches-du-Rhône. Il a mené pendant de longs mois un combat courageux et digne contre la maladie, avec la même détermination qui l'a accompagné toute sa vie.

à laquelle assistaient nombre de personnalités politiques et d'habitants des Bouches-du-Rhône. La ville entière était en deuil. Et c'est aussi dans les rues de cette cité, si chère à son coeur, que les habitants sont venus en masse le long du port lui rendre témoignage de leur affection et de leur reconnaissance, avec émotion, humanité et recueillement. Et les sirènes des bateaux « pleuraient » à l'unisson des coeurs. Le service de l'intérêt général, le don de soi et l'amour du prochain guidèrent sans cesse la vie de Patrick Boré. Né à Toulon le 9 novembre 1956, de parents commerçants, Patrick Boré exerça le beau métier de pharmacien, après des études à la faculté de médecine de Marseille. Installé à La Ciotat,

Engagé en politique depuis les années passées sur les bancs de l'université, il porta la flamme du gaullisme à La Ciotat et s'engagea dans une carrière politique en 1999, en devenant le suppléant du député des Bouches-du-Rhône Bernard Deflesselles. Son élection, en mars 2001, à la mairie de La Ciotat est restée un moment privilégié de sa vie publique.

il s'est consacré à sa ville pendant plus de dix-neuf ans, il l'a transformée et a mis toute son énergie et sa générosité au service des Ciotadens, tant il est vrai qu'un maire est comme un potier qui donne forme à la terre brute. Cette ville lui doit notamment le renouveau des chantiers navals, devenus désormais l'un des fleurons de l'activité de réparation des grands yachts dans le monde, la création du parc du Domaine de la Tour, la rénovation du Port-Vieux ou encore le développement des zones d'activité dédiées aux industries innovantes, sans oublier une politique de l'habitat volontariste permettant aux Ciotadens de vivre et travailler chez eux. Il permit à La Ciotat de renouer avec sa fierté industrielle, mais aussi culturelle, en redonnant vie à l'association La Ciotat Berceau du cinéma, créée pour illustrer la vocation cinématographique de cette ville, liée à la présence des frères Lumière.

Il était profondément gentil et bienveillant, jusqu'au coup d'envoi du match où il se transformait en beau diable. Ce trait de caractère du rugby, il l'avait aussi dans la vie politique : il adorait le combat. » Je le revois, lors Je le revois, lors d'une visite des chantiers, en août 2018, effectuée à son invitation. J'ai en mémoire sa fierté et sa passion lorsque nous parcourions les différentes installations et ateliers, à la rencontre des entreprises entreprises et des salariés du site. Nous avions souligné le succès de la réindustrialisation du chantier naval, et insisté sur l'importance du travail collectif dans cette réussite. Ancré à sa ville, Ancré à sa ville, Patrick Boré l'était aussi à son département. Il fut élu conseiller général du canton de La Ciotat en 2004, réélu en 2011 et 2015, et siégea au total plus de seize années au sein de l'assemblée départementale. Il devint en 2015, aux côtés de la présidente Martine Vassal, premier vice-président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, chargé des relations internationales et européennes, ainsi que des interventions humanitaires. Il fut un élu apprécié de tous, tant au sein de cette assemblée qu'à la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, dont il fut vice-président de 2016 à 2020. En juin 2019, 2019, il s'engagea dans la campagne des élections européennes. Mais notre assemblée l'attirait depuis longtemps. Son arrivée au Sénat, au début du mois d'août 2020, en remplacement de Sophie Joissains, a marqué un tournant dans sa vie. Il mena la liste « Cap sur l'avenir de nos villes et de nos villages lors des élections sénatoriales qui suivirent, aux côtés de nos collègues Valérie Boyer, Stéphane Le Rudulier et Brigitte Devésa, qui lui a maintenant succédé parmi nous. Il fut, comme à son accoutumée, un acteur de rassemblement et d'apaisement. J'ai le souvenir d'une réunion et d'un déjeuner de campagne sénatoriale particulièrement chaleureux, à Aix-en-Provence, en septembre 2020. Il sillonna les Bouches-du-Rhône au cours de cette campagne, allant de mairie en mairie. Élu sénateur, il a gardé la passion de sa ville et de son département. Lorsqu'il passa le flambeau de la mairie de La Ciotat à Arlette Salvo, : « En choisissant le Sénat, je choisis La Ciotat, car je ne quitte pas La Ciotat. [ ...] Avoir deux parlementaires dans un conseil municipal, je crois que c'est important pour une ville aussi.

de « territorialiser » les mesures prises. Il avait ainsi appelé à « réfléchir, en collaboration avec les élus locaux, les fédérations et les organisations professionnelles, à des protocoles sanitaires sûrs et réalisables

du groupe d'amitié France-Arménie, il déposa, en avril 2021, une proposition de résolution par laquelle il invitait le Gouvernement « à exiger de la République d'Azerbaïdjan, sous peine de sanctions, [ ...] la libération sans délai des prisonniers civils et militaires qu'elle détient toujours et la restitution immédiate des corps des soldats arméniens tués au combat ». Ces mots parlent aux présidents des groupes qui m'ont accompagné, un 24 avril 2021, en Arménie.

», « face aux multiples exactions commises par la Turquie et ses alliés, notamment à l'encontre de l'Arménie ». Il fut aussi membre du groupe France-Saint-Siège.

de jeunes migrants érythréens. Ses convictions l'ont toujours porté vers l'autre. Nous garderons de Patrick Boré le souvenir d'un sénateur chaleureux,

J'informe le Sénat que le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants a fait connaître à la présidence le nom du candidat qu'il propose pour remplacer, en qualité de secrétaire du Sénat, Mme Patricia Schillinger, qui a démissionné de cette fonction à compter du 1 octobre 2021. La candidature de M. Dominique Théophile a été publiée et la désignation aura lieu conformément à l'article 2 du règlement. J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication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 J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs est parvenue à l'adoption d'un texte commun.

Dans la discussion générale, la parole est à M. Bruno Retailleau, auteur de la proposition de résolution.

que sept Français sur dix de confession juive disaient avoir fait l'objet d'un acte antisémite : sept sur dix, mes chers collègues ! ... Oui, désormais, de nouveau, la question de l'antisémitisme se pose en France. Mais elle se pose d'une façon radicalement renouvelée.

un autre écosystème s'est mis en place, dans des territoires perdus de la République, gagnés par l'islamisme, des territoires où l'on ne peut plus enseigner la Shoah des territoires où trop souvent nos compatriotes de confession juive se voient cracher au visage les mots de « sale juif »- aujourd'hui, au XXI siècle Dans ces territoires, dans nos écoles publiques, nos écoles de la République, combien reste-t-il d'élèves de confession juive ? Combien de familles ont dû s'exiler, la peur au ventre ?

: désormais, les coupables s'affichent comme des victimes au motif qu'ils appartiendraient à des groupes de « dominés », des groupes de déshérités. Mes chers collègues, hier comme aujourd'hui, un antisémite est un antisémite. Et face à l'antisémitisme, nous ne devons rien céder. Ne rien céder, c'est aussi

l'antisionisme. En tout cas, elle est beaucoup moins nette que certains ne voudraient le faire accroire. Si cette définition est conçue pour être assez large, elle doit être aussi suffisamment stricte pour ne pas blesser la liberté d'opinion : on a le droit, dans notre pays comme dans toutes les démocraties, de critiquer la politique d'Israël,

pour nos compatriotes de confession juive ; c'est une résolution pour la France. Les actes antisémites sont bien sûr des actes dirigés contre des Français en particulier ; mais ils sont d'abord et avant tout dirigés contre la République française, contre ce que nous sommes, contre notre histoire, contre notre projet civique, contre l'essence même de notre beau pays, la France. La parole est à M. Hervé

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues,

Après un nettoyage, cette même stèle sera de nouveau souillée trois jours plus tard. Durant le mois d'août 2021, elle sera abîmée à quatre reprises. Ces actes inacceptables ne sont pas isolés et j'aurais pu, comme vient de le faire mon ami Bruno Retailleau, multiplier les exemples dans tous nos départements ... Si de tels de tels actes se font sous le couvert de l'anonymat, nous assistons également à la résurgence d'un antisémitisme de plus en plus décomplexé, parfois même pratiqué à visage découvert. En témoignent certaines pancartes aperçues cet été dans des manifestations anti-passe sanitaire. L'antisémitisme s'exprime dans la rue, sur les murs des lieux de culte et dans nos cimetières, mais aussi, beaucoup, sur les réseaux sociaux. Pour des milliers de Français, il se traduit par des injures, des intimidations, des discriminations. Comment accepter qu'en France, en 2021, des élèves soient contraints de quitter leur école en raison de leur religion ? Depuis les années 1970, l'opinion publique paraissait pourtant globalement vaccinée contre l'antisémitisme, en France et dans le monde. Mais peu à peu a émergé un nouvel antisémitisme qui, protéiforme, prend souvent pour prétexte la situation au Proche-Orient pour condamner non seulement les Israéliens, mais aussi, sur cette base, un « lobby juif » auquel sont assimilés les juifs de France. Les chiffres du ministère de l'intérieur l'attestent : en 2019, pas moins de 687 faits antisémites ont été comptabilisés par les services de police, ce qui représente une hausse de 27 % par rapport à l'année 2018,

tue : Mireille Knoll, Sarah Halimi, les victimes de l'Hyper Cacher, les enfants de l'école Ozar Hatorah de Toulouse, Ilan Halimi, autant de noms et de visages dans nos consciences, des femmes, des hommes et des enfants sauvagement arrachés à l'affection des leurs par une violence et une haine barbares. on la pensait d'un autre temps. Par son caractère violent et meurtrier, cette nouvelle haine antisémite, apparue dans les années 2000, est sans précédent. Depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais en France on n'avait assassiné des juifs, encore moins des enfants, du seul fait de leur religion. En 1990, la loi tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, dite loi Gayssot, a condamné la négation des crimes contre l'humanité, preuve de l'engagement de la France dans ce combat qui l'honore. Depuis, de nombreux plans interministériels ou nationaux sont venus compléter cette loi. Le dernier en date couvrait les années 2018 à 2020. Cet antisémitisme, né au XX siècle et avançant la plupart du temps sous le masque de l'antisionisme, ne saurait nous laisser indifférents ou démunis. Nous devons le décrire, le définir, le caractériser pour mieux le dénoncer ; c'est là tout le but de la définition proposée par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, organisation intergouvernementale à laquelle appartient la France, comme la quasi-totalité des pays de l'Union européenne.

Je remercie tous mes collègues signataires de cette proposition de résolution pour leur engagement. Il ne s'agit pas non plus d'empêcher toute critique de l'État d'Israël. L'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste le précise d'ailleurs dans ses travaux, indiquant que « critiquer Israël comme on critiquerait tout autre ne peut pas être considéré comme de l'antisémitisme ». La définition que nous vous soumettons a par ailleurs été adoptée par de nombreux pays, dont la France, et par plusieurs villes importantes, comme Paris ou Nice. Elle le fut également par le Parlement européen au printemps 2017. Réaffirmer dans cet hémicycle notre attachement à cette lutte essentielle pour le bien vivre ensemble relève d'une nécessité impérieuse au moment où certains cherchent à réhabiliter le pétainisme et dénient aux enfants tués à Toulouse le droit d'être enterrés en Israël. Parce qu'on ne construit pas une société sûre, pacifique et solidaire sur la haine de l'autre, c'est l'honneur du Sénat que d'adopter cette proposition de résolution.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la période que nous vivons est particulièrement violente et anxiogène pour tous les citoyens de notre pays. Les actes racistes et les actes dirigés contre la communauté musulmane se sont multipliés de façon alarmante ils deviennent des faits divers ; ils ne nous révoltent plus, ou presque plus. Quant aux actes antisémites, forme la plus ignoble du racisme, ils se multiplient eux aussi, et nous inquiètent. Ils inquiètent la communauté nationale, car ils sont une atteinte aux valeurs de la République. République. Je suis petite-fille de déportés ; mon père s'est échappé du Vel d'Hiv grâce à un gendarme français qui a eu pitié de ma grand-mère et a ainsi épargné son fils ... mon père. Penser qu'en France, en 2021, on peut attaquer des personnes au seul motif qu'elles sont juives, et tuer des enfants pour les mêmes motifs, me glace le sang. Penser que certains abrutis utilisent les symboles de la Shoah pour manifester contre le passe sanitaire me donne la nausée. Comment expliquer que certains osent utiliser l'étoile jaune « porte-malheur » ? Comment expliquer à nos parents, qui l'ont portée, ces dérapages insupportables ? Penser que certains

Penser qu'en 2021, en France, terre des Lumières, de l'émancipation des juifs, il faut que nos synagogues soient gardées jour et nuit et que les gardes soient doublées les jours de fête, au point que ma fille a peur d'y emmener ses enfants, me désespère ; et je ne vois pas comment nous inverserons la tendance, madame la ministre. C'est pourquoi je remercie le Gouvernement et le ministre de l'intérieur pour les mesures de sécurité qu'ils consacrent à la protection des lieux de culte-

« Quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous ». Cette citation de Frantz Fanon sonne comme un rappel : le combat contre l'antisémitisme est un combat permanent, un combat pour nous, pour nos enfants et pour nos compatriotes de confession juive, qui font évidemment partie intégrante de la communauté nationale et méritent le même respect que les autres. Hélas, Mireille Knoll, Sarah Halimi, les victimes de l'Hyper Cacher et bien d'autres nous rappellent qu'aujourd'hui, en France, l'antisémitisme est un fléau tenace. La population juive suscite encore des fantasmes, des préjugés, qui conduisent certains à commettre l'irréparable par haine ou simplement par bêtise. Si, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on pouvait légitimement penser que le pire était derrière nous, l'antisémitisme est encore prégnant. L'augmentation de 27 % des actes de ce type en 2019 en témoigne. Ce chiffre doit être cité pour objectiver la haine visible en un Mais il y a aussi ce que l'on ne voit pas, parce que certains ne portent pas plainte ou simplement parce que l'on s'y est habitué, par mithridatisation des esprits. Ce peut-être une phrase, une remarque ou un sous-entendu stigmatisant- autant d'éléments qui chaque jour nous rappellent que l'antisémitisme reste une réalité à combattre, car il est en mutation. Cette proposition de résolution retient la définition suivante : « L'antisémitisme est une certaine perception des Juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard. Les manifestations rhétoriques et physiques de l'antisémitisme visent des individus juifs ou non et/ou leurs biens, des institutions communautaires et des lieux de culte. Cette définition promue par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, approuvée par le Président de la République et par l'Assemblée nationale en 2019, fait débat. Si nous sommes tous d'accord sur le regain que connaît en France sur le fait que nombreux sont les antisémites qui se drapent derrière les drapeaux de l'antisionisme, nous ne devons pas occulter que la définition qui nous est proposée ne fait pas consensus, à l'Assemblée nationale notamment, mais aussi et y compris parmi les intellectuels juifs. Le RDSE n'a pas de position de principe sur ce sujet, sinon celle qui consiste à observer l'étendue du droit existant et les effets qu'engendrerait l'adoption de cette proposition de résolution. Force est de constater qu'entre la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, la loi Gayssot et, surtout, la réforme du code pénal de 1992, qui a aggravé les sanctions en la matière, notre ordre juridique offre une réponse pénale suffisante et complète face aux actes racistes et xénophobes, qui plus est antisémites.

Conscients que cette proposition de résolution est avant tout symbolique et souhaitant réaffirmer leur attachement à la lutte contre toutes les formes de discrimination, les membres du RDSE voteront cette proposition de résolution. La parole

De fait, les préjugés antijuifs perdurent en se renouvelant : juifs riches et assoiffés de pouvoir, juifs responsables de tous les maux, covid compris ... Les pancartes brandies par certains « antivax » et « anti-passe » rappellent les accusations médiévales dirigées contre les juifs propagateurs de la peste » et « empoisonneurs de puits ». Notre lutte contre l'antisémitisme ne doit laisser place à aucune ambiguïté. Pourquoi, dès lors, isoler le phénomène en focalisant l'attention sur la critique d'Israël ? En 2015, au lendemain de l'offensive meurtrière contre Gaza, M. Netanyahou se lance dans la promotion d'une idée simple : « antisionisme égale antisémitisme.

Non contraignante sur le plan juridique, elle demeure un outil de propagande et d'intimidation. En témoignent les pressions exercées par les lobbies pro-israéliens pour la faire adopter par le plus grand nombre possible de municipalités, de partis, d'États. Le 16 juillet 2017, à la fin de son discours prononcé lors de la cérémonie en mémoire de la rafle du Vel d'Hiv, Emmanuel Macron déclarait : « Nous ne céderons rien à l'antisionisme, car c'est la forme réinventée de l'antisémitisme.

Le mot « antisionisme » n'apparaît heureusement pas dans l'exposé des motifs. La définition de l'IHRA me semble pourtant insuffisante et peu éclairante pour qui veut en faire usage. Je voterai de résolution, mais j'aurais préféré que soit retenue la déclaration de Jérusalem, élaborée par des universitaires et approuvée par des centaines de spécialistes de l'histoire des juifs et de l'antisémitisme dans le monde.

La lutte contre l'antisémitisme est un de ces combats, malheureusement toujours d'actualité. Nos sociétés occidentales connaissent le poison d'un antisémitisme qui s'y est enraciné durant des siècles, jusqu'à devenir un préjugé ancré. Cet antisémitisme pluriséculaire, nos sociétés ont choisi de le combattre sans relâche depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, au lendemain de la Shoah. Notre combat, c'est la condamnation de tous les appels à la haine et à l'oubli de la souffrance endurée par les juifs parce que juifs. Je veux ici saluer les paroles prononcées par le président Jacques Chirac lors de son discours historique du 16 juillet 1995, à l'occasion des cérémonies commémorant la rafle des 16 et 17 juillet 1942. Il reconnaissait ce jour-là la responsabilité du régime de Vichy et l'acte « irréparable »- ce sont ses mots - accompli par la France avec la rafle du Vel d'Hiv. Jacques Chirac, par ce discours, a grandi la France. Nous ne pouvons que l'en remercier. Aussi, quand j'entends certains, parfois élus de la République, courir après un polémiste révisionniste ou refuser de le condamner, j'ai mal à ma France.

Qu'ils viennent de l'extrême droite, de la sphère complotiste ou du totalitarisme islamiste, toute parole et tout acte antisémites sont à condamner et à combattre.

de termes, « lutte », « toutes les formes » et « antisémitisme », pris individuellement ou globalement, ont leur importance. Ma famille politique a dans son ADN la lutte contre le racisme et l'antisémitisme ; elle votera donc évidemment cette proposition

où, le 5 octobre 1940, le régime collaborationniste de Pétain transformait un sanatorium en camp d'internement. Près de 1 500 enfants, femmes et hommes y furent internés jusqu'à sa fermeture le 15 septembre 1942, le 15 septembre 1942, avant d'être déportés dans les camps d'extermination de Ravensbrück et d'Auschwitz. Peu d'entre eux survécurent à la barbarie nazie. J'étais également, le 30 novembre 2015, à Sarcelles, nous avons inauguré, en présence de Bernard Cazeneuve, ministre de l'intérieur de l'époque, une place et une stèle en hommage à Yohan Cohen, assassiné à 20 ans, assassiné parce que juif, par un terroriste dans l'attentat de l'Hyper Cacher. Je me souviendrai toute ma vie de la douleur, des visages et des mots de la famille et des amis de Yohan Cohen. Je ne reprendrai pas ici la longue liste des crimes antisémites qu'a connus la France ces dernières années- d'autres l'ont fait avant moi.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je salue à mon tour l'inscription à l'ordre du jour de la Haute Assemblée de ce débat sur la lutte contre toutes les formes d'antisémitisme. L'antisémitisme est un poison, une attaque intolérable contre notre société dans sa globalité, contre le vivre-ensemble et le « faire société Chaque fois que l'antisémitisme frappe, c'est l'égalité entre les citoyens qui est affaiblie. Je ne rappellerai pas l'ensemble des chiffres témoignant de la recrudescence des actes antisémites

selon un sondage conduit par l'IFOP en janvier 2020 ; selon cette même étude, 54 % des agressions verbales se déroulent en milieu scolaire. Ces chiffres inacceptables me donnent le vertige. Nous attendons des écoles et des universités qu'elles soient des lieux d'apprentissage de la vie, de découverte des valeurs humanistes, de tolérance et d'ouverture sur le monde, et non l'occasion pour nos enfants de vivre ou d'être témoins de telles démonstrations de haine. Ces chiffres en disent long sur ce poison qui touche notre jeunesse, qui n'en d'ailleurs pas la seule victime. De tels actes imposent non seulement une condamnation ferme et claire de la part des responsables politiques, mais surtout une action rapide et déterminée pour que cela cesse.

avons vécu, sous prétexte d'une opposition à des mesures sanitaires, un regain de haine inédit en France. Comme vous tous, mes chers collègues, j'ai été profondément choquée de voir défiler un tel antisémitisme antisémitisme décomplexé, assumé à visage découvert, lors de manifestations où des comparaisons abjectes entre le passe sanitaire et l'étoile jaune ont été mises en scène. L'indifférence des personnes qui ont défilé aux côtés de telles pancartes haineuses est inacceptable.

L'indifférence n'est pas un début, c'est une fin. Et, par conséquent, l'indifférence est toujours l'amie de l'ennemi, car elle profite à l'agresseur- jamais à sa victime, dont la douleur est amplifiée quand elle se sent oubliée. J'ai l'espoir qu'un sursaut de conscience puisse avoir lieu dans notre société, car l'antisémitisme n'est pas le problème de nos concitoyens de confession juive : c'est le problème de notre société tout entière. Nous ne devons jamais cesser de combattre tant l'antisémitisme que l'indifférence à tous les instants passe par la répression, l'interdiction, le rappel de la loi par la puissance publique contre ce délit pénal ; mais il passe aussi par une responsabilité collective de chacun des citoyens fermement de tels actes et réagir immédiatement quand ils en sont les témoins. Enfin, ce combat passe par la promotion de l'enseignement de la Shoah, de la mémoire et par une meilleure identification des actes antisémites. À cet effet, notre groupe tient à saluer le travail mené par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste dont la France est membre. Le 26 mai 2016, cette organisation intergouvernementale a adopté par consensus une définition dite « de travail » de l'antisémitisme. Cette définition, qui n'est pas juridiquement contraignante et n'a pas vocation à l'être,

que ces actes passent par des discours de forme visuelle, des stéréotypes ou encore des théories conspirationnistes. D'ailleurs, cette définition tend à garantir la liberté d'expression. Elle ne vise pas à empêcher les critiques à l'égard d'Israël qui sont comparables à celles exprimées à l'encontre d'autres pays. Le groupe RDPI se félicite que le Président de la République ait fait le choix d'endosser la définition de travail de l'antisémitisme

Cette proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui invite le Gouvernement, dans un travail de pédagogie, à diffuser cette définition auprès des services éducatifs, répressifs et judiciaires. Notre groupe soutient une telle perspective, car nous sommes nous aussi convaincus qu'en matière de prévention, d'éducation, de formation ou de répression cette définition constituera un instrument utile pour mieux lutter contre l'antisémitisme. Comme l'a souligné le Président de la République, il ne s'agit pas de modifier le code pénal, encore moins d'empêcher ceux qui veulent critiquer, mais il s'agit de préciser et de raffermir les pratiques de nos forces de l'ordre, de nos magistrats et de nos enseignants dans cette lutte. Par conséquent, le groupe RDPI votera en faveur de cette proposition de résolution, qui respecte les jalons posés par le président Macron. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en guise de préambule, je voudrais relever que l'examen de cette résolution pour lutter contre toutes les formes d'antisémitisme coïncide ce jour avec une cérémonie internationale officielle commémorative de l'Holocauste de Babi Yar à Kiev, en présence du président allemand Frank-Walter Steinmeier et du président israélien Isaac Herzog.

ont été exécutés par balles les 29 et 30 septembre 1941 à Babi Yar, un ravin aux abords de Kiev creusé par une rivière, lieu d'extermination par les nazis de la population juive de la ville dans sa totalité. Il s'agit, mes chers collègues, du plus grand massacre de la Shoah ukrainienne ; il est important de le rappeler en mémoire de tous ces innocents assassinés au nom d'une idéologie barbare. Nous aurions pu marquer aujourd'hui un moment de silence ... Il est intolérable de songer qu'en Ukraine le bataillon néonazi Azov parade en toute liberté avec un symbole qui ressemble particulièrement à celui de la deuxième division SS. La La proposition de résolution de nos collègues Bruno Retailleau et Hervé Marseille est particulièrement à propos ; elle est pertinente et bienvenue. Depuis de nombreuses années déjà, notre pays doit malheureusement affronter une résurgence de l'antisémitisme, comme nous l'avons tous rappelé, et nous déplorons la spirale insupportable d'actes antisémites de plus en plus violents. C'est inédit depuis la Seconde Guerre mondiale. Mireille Knoll, Sarah Halimi, llan Halimi, les victimes de l'école Ozar Hatorah de Toulouse ou encore celles de l'Hyper Cacher de la porte de Vincennes : la liste ne cesse de s'allonger. Ces hommes, ces femmes et ces enfants sont morts parce qu'ils étaient juifs. À ces crimes, il faut ajouter les profanations et dégradations de sépultures et de lieux de culte, les insultes et les agressions physiques. L'antisémitisme, c'est l'intolérance, la haine et la violence. L'antisémitisme, c'est le refus de nos lois. C'est un poison portant atteinte à la France et à nos valeurs républicaines. Il faut le réaffirmer autant que nécessaire, car « il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme même perverse. C'est d'avoir une âme habituée ». Ces mots de Charles Péguy devraient inviter certains candidats à l'élection présidentielle à davantage de modération. Oui, nous avons le devoir d'empêcher que l'inacceptable ne devienne ordinaire, que l'insupportable ne se banalise ! À cet égard, la proposition de résolution vise à faire approuver la définition de l'antisémitisme fixée par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Cette organisation internationale, fondée en 1998, regroupant trente et un pays et à laquelle appartient renforce et promeut l'enseignement de la Shoah, la recherche et la mémoire. La courte définition par l'IHRA est complétée par une série d'exemples afin de permettre de mieux identifier les actes antisémites. La formulation de ces exemples permet de ne pas se heurter à la liberté d'expression. Je félicite les rédacteurs qui précisent que « les critiques à l'égard d'Israël comparables à celles exprimées à l'encontre d'autres pays ne peuvent être qualifiées d'antisémites En effet, la France a toujours considéré les libertés d'expression et d'opinion comme des valeurs les plus fondamentales de la République. Madame la ministre, mes chers collègues, cette définition, qui n'est juridiquement pas contraignante et n'est pas destinée à le devenir, tend à faire connaître et comprendre ce qu'est l'antisémitisme, qu'à apporter un éclairage opportun sur le « fait antisémite ». Elle vise donc notamment les milieux scolaires et universitaires. Elle sera également utile pour les forces de l'ordre et les magistrats. Adopter cette proposition de résolution constitue donc un geste symbolique fort au sein de notre assemblée : c'est montrer notre détermination collective à combattre l'antisémitisme et, par là même, tous ceux qui, par leurs propos ou leurs actes, sèment la haine et l'intolérance. La

! Je le dis au groupe CRCE, le premier texte fort a été la loi Gayssot. Puis il y a eu toute une série de textes, toute une série d'appels, toute une série d'instructions, de circulaires, de décrets

les séides d'une extrême droite néonazie ; protéiforme pour les négationnistes classiques qui font de Pétain le protecteur des juifs français.

Il faut passer à l'acte. Il faut que les réseaux sociaux soient sévèrement punis lorsqu'ils laissent déborder la haine antisémite,

le garant de l'unité de la Nation, de la démocratie et de la République ! Si nous laissons continuer cette progression des actes antisémites, nous remettons en cause la République, la démocratie et la Nation Il n'y a pas de nation sans unité ; il n'y a pas de nation sans autorité de l'État ; il n'y a pas de nation sans un schéma commun, une volonté commune et un destin commun. Voter cette résolution, c'est dire oui à la Nation

madame la ministre, chers collègues, celui qui ne connaît pas son passé est condamné à le revivre. À une époque comme la nôtre, où certains révisent de manière répétée et nauséabonde l'histoire de notre pays et le rôle de Vichy dans les déportations des « juifs français », faut-il que nous discutions d'une résolution sur la définition de l'antisémitisme Bien sûr, il est de notre rôle de légiférer de manière ferme sur ces incriminations pénales, mais ce n'est pas à un Parlement de définir les notions qui font l'objet d'un débat historiographique et de centaines de travaux critiques. nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) et tant d'autres dans le monde, qui parle d'une « certaine perception des Juifs », est loin d'être une référence indiscutable. D'un point de vue très factuel, la résolution présentée exprime le voeu de s'appuyer sur « la définition, non contraignante, de l'antisémitisme fixée par l'IHRA Bien sûr, cela va de soi, nous condamnons tous ici toutes les formes d'antisémitisme. L'antisémitisme, consiste avant tout à ramener quelqu'un à son identité juive, réelle ou supposée, à le caractériser par cette appartenance. C'est une discrimination, un préjugé, une hostilité ou une violence à l'encontre des juifs en tant que juifs. Tout cela est bien antécédent à l'existence même de l'État d'Israël, voire au développement du sionisme. Le sujet est grave, il est dramatique. Il appelle d'autant plus à la nuance. Chacun, sur nos travées, condamne de manière forte et sans réserve la montée des actes de violence envers les juifs, ainsi que la haine exprimée par certains envers ceux qu'ils estiment responsables de leur malheur ou qu'ils imaginent contrôlant des zones entières de notre société. L'antisémitisme évolue, surtout ses formes, ses raisons supposées, ses justifications inacceptables et toujours empreintes de mauvaise foi. Le révisionnisme, qui vient parfois de la droite et de l'extrême droite, est un antisémitisme qui s'exprime sous la forme de profanation de cimetières et de synagogue. Il faut le combattre. L'écho que certains donnent à de trop nombreuses théories complotistes sur la pandémie et le développement abject des pancartes « Qui ? » n'arrangent rien. Tout cela doit être combattu. Quels que soient les chiffres, nous devons lutter Cette haine aveugle, cette révision de l'histoire à des fins démagogiques n'ont pas de place dans notre république. Les défenseurs de cette résolution et de cette définition de l'antisémitisme y voient la possibilité de qualifier d'antisémites les attaques antisionistes motivées par une haine des juifs. Pourtant, rien dans la définition même proposée par l'IHRA ne parle de sionisme ou d'antisionisme. Ce sont les exemples publiés dans la déclaration de 2016 qui évoquent les conditions dans lesquelles la critique d'Israël pourrait être antisémite. Et c'est bien sur ce point que nous nous devons être vigilants, nuancés, sans que cela remette en cause notre volonté de combattre de manière pleine et entière toutes les formes d'antisémitisme. Le Président de la République a déclaré vouloir élargir la définition de l'antisémitisme à l'antisionisme. Je sais que les auteurs de la résolution aiment à rappeler que l'IHRA a affirmé qu'« une critique d'Israël similaire à celle portée contre n'importe quel autre pays ne peut être vue comme antisémite Mais c'est bien parce que cela n'est pas si clair dans les définitions et les exemples qui ont été retenus que l'IHRA, puis vous-mêmes, à l'alinéa 7, estimez nécessaire de vous dédouaner de cette interprétation.

Si l'on peut considérer qu'il existe dans certaines attaques formulées contre Israël des dérives antisémites, les critiques de la politique des gouvernements israéliens ne peuvent y être assimilées sans nuire au combat contre l'antisémitisme et le racisme. Nous refuserons toujours cette instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme. Une tribune parue dans et signée par des personnalités juives concluait : « Nos opinions sur le sionisme peuvent être diverses, mais nous pensons tous, y compris ceux qui se considèrent comme sionistes, que cet amalgame est fondamentalement faux. » Mes chers collègues, oui l'antisionisme est parfois le faux nez de l'antisémitisme, mais le simple fait qu'il puisse servir d'alibi à ce nouvel âge de l'antisémitisme ne doit pas justifier que nous cédions en validant ce faux-semblant. Le droit pénal est d'interprétation stricte, mais les juges ne sont pas des robots et ils sont là pour évaluer la situation. L'arsenal juridique est déjà important pour sanctionner l'antisémitisme. Attaquer une personne du fait de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, à une nation, à une race ou à une religion déterminée est déjà sanctionné. Cela fait l'honneur de notre République et de notre Constitution.

sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. On

Monsieur le président, chers collègues, la haine du juif en France, c'est l'histoire longue de deux mille ans de mesures d'éloignement, de législations d'exclusion, d'accusations criminelles, de persécutions, de pogroms et de génocides. Dans sa monumentale, Léon Poliakov montre que cette haine du juif trouve son origine dans l'Antiquité puis se renouvelle dans la constitution du corpus théologique et politique du christianisme naissant. Je le cite, « pour l'économie du christianisme, il fallait dorénavant que les juifs fussent un peuple criminellement coupable ». Reconnaissons-le, chers collègues, l'antijudaïsme a participé de la formation d'une certaine identité chrétienne de l'Occident. Ainsi, en 1096, les croisés massacrent les juifs de Rouen. La deuxième croisade de 1146 est précédée des mêmes pogroms et l'abbé Pierre de Cluny les justifie ainsi : « À À quoi bon s'en aller au bout du monde, [ ...] pour combattre les Sarrasins, quand nous laissons demeurer parmi nous d'autres infidèles qui sont mille fois plus coupables envers le Christ que les mahométans ? Il existe un antijudaïsme d'État aussi ancien dont l'histoire est marquée par les édits d'expulsion des juifs de Childebert en 533, de Dagobert en 633, de Philippe Auguste en 1182, de Saint Louis en 1254, de Philippe le Bel en 1306 et de Charles VI en 1394. Il faut ajouter à cette terrible série les mesures prises par Napoléon Bonaparte, au moment du Concordat, pour interdire aux juifs de s'installer en Alsace. Il les justifiait par sa volonté « d'atténuer, sinon de guérir la tendance du peuple Juif à un si grand nombre de pratiques contraires à la civilisation et au bon ordre de la société ». Ce qui est désigné dans ce projet de résolution par l'expression « antisémitisme contemporain » s'inscrit fondamentalement dans l'histoire trop longue d'un antijudaïsme millénaire dont son exposé des motifs ne nous dit malheureusement rien. Ainsi, sans nier l'existence de formes actuelles d'antisémitisme prônant la destruction de l'État d'Israël, comment ne pas reconnaître dans les théories complotistes qui expliquent la covid comme le fruit d'une conspiration juive des résurgences des thèses médiévales qui accusaient les juifs de l'anéantissement de la chrétienté par l'épidémie ? C'est notre première réserve sur ce projet. Notre deuxième objection porte sur le choix de la définition de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, qui est imprécise et dont l'utilisation politique très partisane a été justement dénoncée par Kenneth Stern, l'un de ses rédacteurs. Cette définition n'était qu'une définition de travail. Depuis lors, un groupe de plus de deux cents spécialistes l'a reprise pour en lever les ambiguïtés dans un texte publié en 2020 sous le titre de Déclaration de Jérusalem. est plus pertinente parce qu'elle inscrit les antisémitismes d'hier et d'aujourd'hui dans le même processus idéologique d'assimilation des juifs aux forces du mal. Cette déclaration rappelle avec force que « le combat contre l'antisémitisme ne saurait être dissocié de la lutte globale contre toutes les formes de discrimination raciale, ethnique, culturelle, religieuse et sexuelle Enfin, nous regrettons vivement qu'une résolution citant l'Alliance pour la mémoire de l'Holocauste ne mentionne aucunement la nouvelle irruption dans le débat public de thèses négationnistes et de tentatives de réhabilitation de l'État français du maréchal Pétain. Très Souvenons-nous de la déclaration, au nom de la France, du président Jacques Chirac, le 16 juillet 1995, lors de la commémoration de la grande rafle de juillet 1942 : « La folie criminelle de l'occupant a été secondée par des Français, par l'État français, [ patrie des Lumières et des droits de l'homme, terre d'accueil et d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bourreaux. Je le cite toujours : « Transmettre la mémoire du peuple juif, des souffrances et des camps. [ ...] Reconnaître les fautes du passé, et les fautes commises par l'État. Ne rien occulter des heures sombres de notre histoire, c'est tout simplement défendre une idée de l'homme, de sa liberté et de sa dignité. C'est lutter contre les forces obscures, sans cesse à l'oeuvre. » Cette déclaration nous honore, nous oblige Elle impose au Sénat d'éclairer davantage nos concitoyens sur les deux mille ans de cet antijudaïsme qui aboutit à l'inhumanité absolue de la Shoah. Engageons, chers collègues, ensemble, dans l'unité, ce travail de fond à partir de la Déclaration de Jérusalem. La parole

Qu'est-ce donc que la haine ? Aucune définition dans aucun dictionnaire du monde ne satisfera tout à fait notre volonté de comprendre. Notre besoin de consolation, face aux effets désespérants de la haine, restera à jamais inassouvi, mais nous savons qu'elle laisse dans son affreux sillage des images imparables qui marquent au fer rouge nos imaginations et nos consciences meurtries. Ces images de la haine en action habitent nos mémoires au point de nous hanter parfois sans qu'on puisse leur échapper. Vous me permettrez d'évoquer devant vous, deux de ces images sorties tout droit de l'album souvenir de l'horreur antisémite. Voici la première : Toulouse, 19 mars 2012, huit heures du matin, devant l'école Ozar Hatorah, un petit garçon terrifié rampe dans la rue près du corps de son père et de son frère. Ils viennent d'être abattus par un assassin en scooter équipé d'une caméra. Car il ne suffit pas de tuer, il faut aussi archiver la tuerie, sans doute pour en jouir davantage. Le petit garçon est achevé à son tour. Puis le tueur s'en prend à une fillette qu'il poursuit après l'avoir blessée à l'épaule ; il la saisit par les cheveux et la tue à bout portant. Le père des garçons avait 30 ans ; ses fils 3 ans et 6 ans. La petite fille avait 8 ans. Jonathan, Gabriel et Arié Sandler, ainsi que Myriam Monsonégo : tels étaient leurs noms. Tous coupables d'être juifs aux yeux de leur bourreau. La seconde image est celle-ci : Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne, le 13 février 2006. Un jeune homme est découvert aux abords de la voie ferrée du RER C. Son crâne est tondu, sa bouche bâillonnée, son corps nu est couvert d'ecchymoses et de traces de brûlures. Il a deux entailles à la gorge. Il est à l'agonie. Il meurt. Il avait 23 ans. Ses bourreaux, au nombre d'une vingtaine, l'ont torturé pendant trois semaines parce qu'il était juif. Ilan Halimi était son nom. Des journées entières, des mois, des années, ne suffiraient pas pour feuilleter, crime après crime, l'interminable album souvenir de la haine antisémite. Combien de tortures ? Combien d'actes de barbarie ? Combien de profanations, d'humiliations, d'exils ? Combien de morts ont-elles été perpétrées par cette haine au cours des millénaires ? Y a-t-il une époque, une nation, qui en furent exemptes ? Je ne saurais le dire Aujourd'hui, nous voyons renaître, dans notre propre pays, la bête immonde de l'antisémitisme. Certes, elle ne se manifeste pas toujours sous les aspects atroces que je viens d'évoquer. Il lui arrive même de se camoufler sous des masques qui savent feindre l'innocence. Elle n'en est pas moins redoutable et mortelle. La violence haineuse ne brandit pas toujours des armes létales, mais elle peut aussi tuer par la simple parole. Car la vie et la mort, mes chers collègues, sont au pouvoir des mots. Que dire alors de la peur ? Devant la recrudescence des actes antisémites, face à la multiplication des comportements haineux, des propos discriminants et de leur banalisation, le poison de la peur s'instille dans les consciences au point de pousser certaines personnes à quitter la France. Non, mes chers collègues, ce ne sont pas les juifs inquiets qui doivent fuir la France. C'est la France qui doit tout mettre en oeuvre pour bannir la peur et dénoncer avec clarté la haine antisémite afin de la combattre absolument. Je suis faite pour partager l'amour et non pour partager la haine ! » Cette proclamation d'Antigone, ô combien je voudrais la faire mienne et qu'elle devienne une déclaration de foi en l'humanité ! Devrait-on pour cela inscrire l'empathie au programme de l'éducation nationale ? J'en doute. L'utopie n'est sans doute pas la meilleure réponse à opposer à la violence d'une société, mais que l'on me permette un instant de rêver à une France où le mot antisémite n'aurait plus aucun sens pour personne.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, « heureux comme un juif en France » : pendant très longtemps, c'est par cette locution que les communautés juives d'Europe signifiaient leur admiration pour la France. Le philosophe juif lituanien Emmanuel Levinas citait son grand-père qui répétait en se référant à l'affaire Dreyfus : « Un pays qui se déchire, qui se divise pour sauver l'honneur d'un petit officier juif, c'est un pays où il faut rapidement aller. » L'engagement acharné d'Émile Zola, d'Anatole France, de Georges Clemenceau, de Jean Jaurès et de quelques autres en faveur du capitaine Dreyfus avait fini par traverser les frontières et faire le tour de l'Europe. Ces hommes sauvèrent l'honneur de la France. Ils furent l'honneur de la France. Hélas, cinquante ans après l'affaire Dreyfus, la communauté juive de France allait connaître l'oppression, les persécutions, la déportation et l'extermination. N'en déplaise à celles et à ceux qui essaient de relativiser le rôle du régime de Vichy dans la Shoah, et n'en déplaise à un candidat putatif à la prochaine élection présidentielle, notre référence en la matière reste et restera le discours du 16 juillet 1995 du président Jacques Chirac,

la France et la communauté juive de France furent la cible des attentats terroristes islamistes, meurtriers, de l'école Ozar Hatorah et de l'Hyper Cacher. La France et la communauté juive de France eurent également à déplorer les crimes antisémites perpétrés contre Ilan Halimi, Sarah Halimi, Mireille Knoll. L'antisémitisme, aujourd'hui, ce sont autant des profanations de tombes juives que des souillures sur les synagogues. Ce sont aussi bien les violences physiques que les injures gratuites. Ce sont aussi bien les messages de haine sur le Net que la réécriture révisionniste et négationniste en 2021 de ce drame absolu que fut la Shoah. C'est contre ces préjugés, ces stéréotypes, ces amalgames qu'il nous faut nous élever. Toutes les formes d'antisémitisme sont à combattre, qu'elles viennent de l'extrême droite ou des nébuleuses islamistes. Nous ne faisons pas de distinction, car ces idéologies mortifères se rejoignent dans la haine des juifs. Mes chers collègues, la lutte contre l'antisémitisme doit mobiliser les forces républicaines au Parlement. Nous le faisons une nouvelle fois à l'occasion du vote de cette proposition de résolution. La lutte contre l'antisémitisme doit aussi mobiliser tous les pouvoirs publics, qu'il s'agisse de l'éducation nationale, de la police, de la gendarmerie ou de la justice. Cette mobilisation générale, nous la devons à nos compatriotes de confession juive. Fatigués d'être pris pour cibles, ils sont de plus en plus nombreux à se demander si leurs enfants ont encore leur place dans l'école de République. Ils sont également de plus en plus nombreux à se demander s'ils ont encore un avenir sur le sol de France. Alors, depuis cette tribune, je voudrais dire à ces compatriotes

en fidélité à notre engagement ancien et renouvelé contre l'antisémitisme, le racisme, la xénophobie, l'homophobie et toutes les discriminations qui sont autant de menaces pour notre cohésion nationale et notre pacte républicain. Nous voterons cette proposition de résolution, car nous sommes les héritiers d'une histoire que nous avons eu le courage de regarder en face. Cette histoire faite d'ombres et de lumières, c'est la nôtre. Inspirés par tous ces résistants, célèbres et anonymes, par tous les Justes parmi les nations, dont nous gardons le souvenir ardent, inspirés par la mémoire de ces héros tombés face au péril islamiste, nous vous disons, chers compatriotes de confession et de culture juives, vous n'êtes pas seuls Nous vous le disons, à vous ainsi qu'à toutes les Françaises et à tous les Français, car nous sommes les héritiers d'une histoire et les passeurs d'une mémoire. Nous vous le disons, car nous sommes dépositaires d'une espérance et d'une promesse que la République fait à chacun de ses enfants : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions religieuses. Être conscients de cet héritage moral, être volontaires pour réaliser cette espérance, c'est se hisser à la hauteur de ce que le général de Gaulle appelait « une certaine idée de la France ». La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans le plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme que le Gouvernement a lancé en 2018, Édouard Philippe, alors Premier ministre, a écrit : « Le racisme et l'antisémitisme ont tué en France ces dernières années. Ils s'expriment dans la rue, sur les murs des lieux de culte, sur les réseaux sociaux, dans les forums de discussion. Pour des millions de Français, ils se traduisent par des injures, des intimidations, des coups, des discriminations. Des élèves doivent quitter leur école en raison de leur religion. Vous me direz que les services de l'État mettent en place des politiques en ce sens. Mais quels sont les résultats de ce qui a été entrepris depuis que l'on a fait ce constat terrible ? Qu'avons-nous fait pour ne plus connaître des drames comme ceux, terribles, qui ont sidéré la France ? Ou pour juguler l'antisémitisme « ordinaire », celui qui se libère dans l'espace public, sur internet et les réseaux sociaux et qui fait tellement de dégâts au quotidien En Alsace, région où je suis née, où j'ai grandi, et dont je suis aujourd'hui élue, nous avons un passé historique unique, dense et riche, un passé commun avec la communauté juive, dont la présence est millénaire. Les juifs d'Alsace ont contribué à forger la culture alsacienne. Nous en retrouvons des traces dans notre dialecte empreint de yiddish, dans les chants, dans la littérature, dans la cuisine et le patrimoine bâti.

chassés au XIV siècle, au moment de la Grande Peste noire, accusés d'empoisonner les puits ; spoliés et humiliés en 1848 dans mon village du Sundgau ; éradiqués d'Alsace pendant la Seconde Guerre mondiale de tout temps, et particulièrement lors des périodes de crise, nous avons connu des flambées antijuives, comme partout en France. Mais nous avons toujours eu à coeur de maintenir le « savoir vivre ensemble » spécifique à notre territoire de concordat. Car en Alsace-Moselle, les relations avec les cultes ne sont pas régies par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, mais par le concordat de 1801. Notre concordat a permis de développer une culture du dialogue, un savoir-vivre ensemble fondé sur la compréhension, le respect et l'amitié entre les différentes religions et les autorités « civiles C'est ainsi que nous luttons contre les malentendus et les hostilités séculaires. À la région Grand Est, tout comme à la Collectivité européenne d'Alsace (CEA), les élus sont conscients de la nécessité d'entretenir un dialogue apaisé entre les cultes les affaires religieuses ne sont pas un tabou. Dans chacune des collectivités, des conseillers et des services sont chargés du dialogue interreligieux. Pour autant, l'Alsace n'échappe pas à la poussée antisémite. C'est pourquoi la CEA a soutenu la mise en place d'un dispositif appelé les « veilleurs de mémoire » pour lutter contre les profanations de tombes. Les autres cultes présents sur notre territoire participent à ce dispositif et le font connaître. Déjà 80 bénévoles, de toutes confessions, se sont engagés dans le réseau qui s'est constitué en 2019 avec une douzaine de veilleurs au départ. L'objectif est de leur permettre d'accueillir des collégiens pour témoigner de leur engagement citoyen. Car la lutte contre ces relents antisémites passe nécessairement par la prévention, par l'éducation et par la culture. À ce titre, l'apprentissage de l'histoire est essentiel, et les professeurs ne doivent plus craindre d'aborder certaines périodes en classe, à commencer par la Shoah, dont certains n'osent plus prononcer le nom. La recrudescence des actes antisémites est l'affaire de tous. Et en tant que politiques, notre responsabilité est grande. Notre défi commun est de lutter contre l'indifférence et la banalisation de ces actes, de nous doter d'outils efficaces qui renforceront et protégeront notre nation, ses valeurs morales et politiques. À ce titre, je salue le travail engagé par Bruno Retailleau et Hervé Marseille pour mieux définir ce qu'est l'antisémitisme, et je les en remercie. C'est un premier pas qui, je l'espère, sera suivi d'autres prochainement.

Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, en 2004, le rapport de Jean-Pierre Obin sur les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires nous apprenait que le racisme antijuif avait très nettement supplanté, à l'école, le racisme antimaghrébin. Il mettait en évidence une stupéfiante réalité : les enfants juifs français, et ils sont les seuls dans ce cas, ne peuvent pas être scolarisés dans n'importe quel établissement. Dès lors, si l'antisémitisme prospère dans nos écoles, comment ne pas soupçonner qu'il s'épanouisse encore bien au-delà de leurs murs et qu'il n'ait jamais cessé de diffuser son venin dans notre pays ? À cet égard, les centaines de faits à caractère antisémite recensés chaque année doivent nous rappeler que nos compatriotes de confession juive demeurent ô combien éprouvés ! Et pour cause. Lorsqu'une vitrine est souillée de l'inscription, lorsque le visage de Simone Veil est scarifié d'une croix gammée, lorsque Alain Finkielkraut est lynché verbalement, c'est le fantôme le plus ignoble et le plus diabolique de l'Histoire qui ressurgit. Lorsqu'on poignarde Mireille Knoll, lorsque Mohammed Merah assassine de jeunes enfants de l'école Ozar Hatorah, lorsque l'on profane des tombes juives, parce que juives, c'est la plus insoutenable des résurgences du passé de l'Europe qui nous remplit d'effroi. ce n'est pas de la Nuit de cristal que je vous fais le récit. Je vous parle de Paris en 2019, de Sarre-Union en 2015, de Toulouse en 2012. C'est notre France, notre siècle. Ce fléau qui habite notre civilisation ne s'est pas malheureusement pas éteint à la libération des camps. Les années noires sont certes derrière nous, mais la bête immonde est là, tapie dans l'ombre, mâchoire acérée suintant de haine, prête à bondir et le ventre encore fécond. simplement pris d'autres visages. Celui de la folie islamiste, où la détestation des juifs s'inscrit au coeur d'une dialectique anti-occidentale. Celui aussi d'un antisionisme absolu, qui n'est pas la seule critique, légitime, de la politique d'Israël, mais qui permet de s'adonner à l'antisémitisme le plus décomplexé sans encourir l'opprobre de ressusciter tout un passé d'oppression et de génocide. L'oubli, plus latent, ne nous menace hélas pas moins. Car seul le souvenir est au service de la sagesse, le souvenir comme remède universel à l'égarement de l'homme sur les chemins de la barbarie. L'école est au-devant de cette bataille culturelle. Elle est un haut lieu de transmission des valeurs de la République, sans lesquelles les tragédies d'hier reviendront fatalement sur nos rivages, au gré des vagues de la haine ordinaire. Elle doit, avec ses professeurs, porter inlassablement le souvenir des crimes antisémites. Le devoir de mémoire, de pédagogie et de sagesse doit nous guider, nous éclairer et renvoyer ces démons là où ils doivent rester : dans les marécages de l'indignité absolue.

Souvenons-nous de ce qu'il qualifiait de crime : le crime « d'exploiter le patriotisme pour des oeuvres de haine », « d'empoisonner les petits et les humbles, d'exaspérer les passions de réaction et d'intolérance ». Ces mots sont d'hier, et pourtant ils pourraient être d'aujourd'hui. ne doivent avoir d'autre fin que de nous éveiller à la poursuite de la lutte contre l'antisémitisme qui, comme tous les racismes, n'a pas sa place dans une République dont la devise est « Liberté, Égalité, Fraternité ». Fraternité ». « Les souvenirs sont nos forces. Quand la nuit essaie de revenir, il faut allumer les grandes dates, comme on allume des flambeaux », a écrit Victor Hugo. Ne rendons surtout jamais illisibles les pages les plus sombres de l'histoire de l'humanité, veillons à ce que personne ne puisse jamais les récrire,

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, l'écrivain israélien Amos Oz raconte que son père, lorsqu'il était enfant dans l'Europe de l'entre-deux-guerres, avait découvert un matin, sur le mur en face de sa maison, l'inscription suivante : « Juifs, fuyez au Proche-Orient ! » C'est ce qu'il fit, ajoute Amos Oz. Il quitta l'Europe contaminée par l'antisémitisme et s'installa à Jérusalem. Bien des décennies plus tard, vers la fin du XX siècle, il revint visiter sa ville natale. Sur le même mur était maintenant écrit un autre slogan

un supposé cosmopolitisme ou, au contraire, un excès d'enracinement dans une terre -, c'est la même haine ontologique, la même haine antisémite. Nous devons combattre de toutes nos forces diverses formes de cet antisémitisme. C'est pour cela que nous sommes réunis au sein de la Haute Assemblée. Comme vous, j'aimerais ne pas avoir à parler d'antisémitisme. Mais la réalité est là, est là, récurrente. La réalité, c'est que la haine antisémite connaît une poussée préoccupante dans notre pays depuis deux décennies. Que les actes antisémites vécus au quotidien par nos concitoyens- menaces, injures, dégradations, inscriptions, agressions physiques ... -ont augmenté. Qu'internet, où l'anonymat autorise toutes les outrances, fournit un exutoire et une caisse de résonance à l'antisémitisme. Que des citoyens français ont été tués sur notre territoire parce qu'ils Ilan Halimi, les enfants de l'école Ozar Hatorah de Toulouse et leur professeur, les otages de l'Hyper Cacher de la porte de Vincennes, Sarah Halimi, Mireille Knoll. Tous ont été cités à cette tribune et je veux, à mon tour, leur rendre hommage. La réalité, c'est que plus d'un tiers de nos concitoyens de confession juive se sentent aujourd'hui menacés en raison de leur appartenance religieuse, contre 8 % pour l'ensemble des Français. Que près de la moitié d'entre eux

Ce sont ces listes de personnes supposément ou réellement juives exhibées sur des pancartes, avec ce mot glaçant : « Qui ? » ! Avec la pandémie, un antisémitisme latent s'est aussi révélé au grand jour. jour. La crise sanitaire a réveillé de grandes peurs et ranimé le désir de trouver des boucs émissaires. Elle a fait ressurgir le fantasme, sinistre, d'un supposé complot juif international qui dirigerait le monde. Nous ne pouvons pas accepter le retour de cet antisémitisme décomplexé dans l'espace public, cette manière de désigner les juifs à la vindicte et de leur imputer des crimes imaginaires. C'est ce type de représentations qui prépare et, parfois, tente de justifier le passage à l'acte. L'antisémitisme n'a pas sa place dans ce pays. Nous le combattons avec la plus extrême fermeté. Nous le devons à nos concitoyens de confession juive dont l'histoire, depuis l'Antiquité, est profondément enracinée dans notre territoire et qui ont contribué à façonner le visage et les valeurs de notre pays. Ils ont le droit, comme chaque citoyen, de vivre en paix chez eux. Nous le devons aussi à la Nation tout entière. Comme le rappelait avec force, en décembre 2019, le Président de la République, l'antisémitisme est toujours le signe avant-coureur d'autres formes de haine, quand il n'est pas celui d'une violence de masse. Il nous concerne tous, il concerne la République tout entière. Nous le savons, et vous l'avez dit, il n'est pas possible de mener un combat contre un adversaire que l'on ne connaît pas. L'antisémitisme a beaucoup évolué. Il ressemble en partie seulement à celui que nos manuels d'histoire nous ont appris à identifier. Il continue d'avoir les traits de ce vieil antisémitisme de l'extrême droite européenne, qui accuse les « juifs » d'être des traîtres à la Nation. Mais il est également présent à l'autre extrémité de l'arc politique où, trop souvent, on associe facilement les juifs aux dominants et où l'on en veut à Israël de tout simplement exister. exister. Il prend aussi le visage de l'islamisme radical et de tous ses complices, nous le savons bien. Toutes ces formes d'antisémitisme sont détestables. Nous devons leur livrer bataille sans répit. Parce que l'antisémitisme est ainsi multiforme et complexe, nous avons besoin, pour mieux le combattre, de mieux le définir. C'est la raison pour laquelle la France a décidé, comme le Président de la République l'a annoncé dès 2019, de mettre en oeuvre la définition de l'antisémitisme adoptée par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Cette définition de travail permet d'identifier la variété des motifs qui composent, hélas, l'antisémitisme contemporain : fantasme du complot juif international, statut de bouc émissaire, pouvoir supposé de l'argent, négation de la Shoah, reproche conspirationniste et négationniste fait aux juifs d'avoir inventé ou exagéré ce qu'a été l'Holocauste, mais aussi remise en question du simple droit de l'État d'Israël à exister.

donc pas de valeur juridique contraignante. Elle ne modifie pas notre droit. Les dispositions qui nous permettent de sanctionner l'antisémitisme restent les mêmes : l'injure publique, la diffamation, la provocation à la haine ou à la violence ... Mais cette résolution, même sans force contraignante,

Elle permettra de mieux identifier, de mieux caractériser l'antisémitisme. Le deuxième point, sur lequel je tiens à insister, concerne la critique d'Israël. La résolution précise, et c'est très important, que la définition de l'antisémitisme que nous recommandons n'est pas contradictoire avec la liberté de critiquer les politiques menées par le gouvernement israélien. Nous pouvons continuer à débattre des orientations de cet État, comme on le fait pour les autres pays, et d'autant plus qu'il s'agit d'un État ami de la France. Comment pourrait-il en être autrement ? C'est une chose normale en démocratie que de dire : « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. » C'en est une autre, qui nous fait basculer dans la haine et la violence, que d'affirmer : « Vous n'avez pas le droit d'exister !

Parce que le combat se mène de plus en plus dans l'espace cyber, la plateforme de signalements Pharos fonctionne maintenant sept jours sur sept, et le dialogue avec les acteurs du numérique a été relancé. Un réseau d'enquêteurs et de magistrats formés à la lutte contre la cyberhaine a été mis en place. haineux sur internet, un parquet spécialisé dans le numérique et un observatoire de la haine en ligne ont été créés. Un effort massif de formation a été accompli, notamment- je tiens à le souligner -auprès des policiers et des gendarmes, mais aussi des enseignants et des magistrats. Notre soutien aux institutions mémorielles a été renforcé et amplifié.

Je vous le dis, notre arsenal de mesures pour continuer à lutter sans relâche contre l'antisémitisme sera renforcé dans le cadre du prochain plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme qui sera adopté, je l'espère, Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement soutient pleinement et sans réserve cette résolution. Elle nous apporte un moyen très concret pour lutter avec plus de force contre l'antisémitisme. Elle adresse aussi un message : celui d'une France résolue à agir, d'une France qui ne s'habitue pas à la haine et aux passions mauvaises,

la conférence des présidents a décidé que les interventions des orateurs valaient explication de vote. Je mets aux voix la proposition de résolution. Mes chers

est suspendue. La séance est reprise. Je rappelle au Sénat que le groupe RDPI a présenté la candidature de M. Dominique Théophile en qualité de secrétaire du Sénat. La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai prévu par l'article 2 du règlement. En conséquence, je déclare cette candidature ratifiée et je proclame M. Dominique Théophile secrétaire du Sénat. groupe Les Républicains, l'examen de la proposition de résolution portant sur la nécessité de reconnaître le Gouvernement d'unité nationale de Birmanie, présentée, en application de l'article 34-1 de la Constitution,

à la suite du coup d'État de février dernier, et de proposer une initiative. Je remercie également le président du groupe Les Républicains, Bruno Retailleau, d'avoir accepté d'inscrire ce texte rapidement sur le temps du groupe Les Républicains. Je sais également toute l'attention de M. le président, du Sénat, Gérard Larcher, ainsi que de notre collègue Joëlle Garriaud-Maylam, présidente du groupe d'amitié France-Birmanie. Enfin, je sais gré à tous nos collègues représentant les différents groupes politiques du Sénat- ils sont nombreux -, qui ont accepté de cosigner la présente proposition de résolution. Ce bel élan d'unité et de solidarité démontre à nos amis Birmans, dont certains sont présents en tribune et que je salue, combien le sujet de leur avenir rassemble en France, au-delà des clivages partisans. s'en souvient, les élections nationales de novembre 2020 en Birmanie, il y a donc un an à peine, ont été largement remportées- 83 % des voix avec un taux d'abstention très bas -par la Ligue nationale pour la démocratie. Cette élection porteuse d'espoir traduisait une forte adhésion à la transition démocratique dans laquelle le pays s'est engagé depuis 2015. Quelques mois plus tard, les militaires précédemment au pouvoir ont organisé le 1 février 2021, veille de la rentrée du Parlement, un coup d'État violent afin d'empêcher son installation et de reprendre ainsi les commandes du pays. Ce coup d'État qui s'est accompagné de la proclamation de l'état d'urgence a plongé le pays dans la violence et la terreur. Si certains des élus « légitimes », issus démocratiquement des urnes, ont pu s'enfuir, d'autres ont été faits prisonniers par la junte. À travers la totalité du pays, la population s'est immédiatement soulevée en appelant à la désobéissance civile et à des manifestations pacifiques- au début -contre le pouvoir militaire, dont la réaction a été de réprimer en arrêtant, en torturant et en tuant des civils. En plus des personnalités politiques, de nombreux défenseurs des droits de l'homme, journalistes, membres de la société civile, universitaires, enseignants, personnels médicaux, chefs religieux et ressortissants étrangers ont été arrêtés et restent pour la plupart détenus arbitrairement par l'armée birmane.

c'est toute la raison d'être de cette proposition de résolution : inviter le Gouvernement français à procéder à une reconnaissance du Gouvernement d'unité nationale de Birmanie.

de l'Asie du Sud-Est) du 24 avril 2021 s'est conclu par un consensus sur cinq points : la nécessité immédiate de mettre fin aux violences, l'ouverture d'un dialogue constructif entre toutes les parties concernées, la désignation d'un envoyé spécial de la présidence de l'Asean pour faciliter la médiation du processus de dialogue, l'aide humanitaire, et enfin la visite en Birmanie de l'envoyé spécial, lequel n'est pour l'heure pas autorisé par les autorités militaires à entrer sur le territoire birman, pas rencontrer toutes les parties prenantes, notamment les personnalités emprisonnées. Il en est de même, d'ailleurs, pour l'envoyé de l'ONU. Les ministres des affaires étrangères des pays du G7 ont rappelé que les personnes responsables de violations du droit international aux droits de l'homme devront rendre des comptes. Au cours des derniers mois, trois séries de sanctions ont été prises par l'Union européenne à l'encontre des responsables de ce coup d'État et des intérêts économiques des forces armées birmanes.

En ciblant tant les avoirs que les secteurs des pierres précieuses et du bois, ces mesures visent à limiter la capacité de la junte à tirer profit des ressources naturelles du pays. Quant à l'embargo sur les armes et les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression, il reste en vigueur. En revanche, la question des revenus pétroliers n'est pas résolue de manière satisfaisante, alors que la population manque cruellement de tout. La pression financière sur les membres de la junte devrait être accrue. Mes chers collègues, le temps presse, car la situation n'évolue guère favorablement. Elle pourrait progressivement prendre le tour d'une guerre civile marquée par une répression sévère des autorités militaires, d'autant plus que toutes les grandes ethnies participent au Gouvernement d'unité nationale. Les civils en viennent à s'armer et à s'organiser en groupes de défense, sans pour autant disposer de la formation contrairement aux forces de sécurité. Ils lancent désormais des actions de sabotage. Le week-end dernier a ainsi été marqué par de nombreuses violences. Depuis février, le bilan de cette crise politique est lourd. Selon certaines estimations, 1 120 civils- en réalité certainement beaucoup plus -ont été tués. Nombre d'entre eux sont morts en prison à la suite de tortures. Au moins 6 700 personnes ont été arrêtées. Leurs familles ne savent ni où elles se trouvent ni même si elles sont encore en vie. Parmi eux, des anonymes, des médecins, des infirmières, des journalistes, des artistes. De nombreux enfants et femmes enceintes ont été assassinés, des enfants ont été enlevés puis défigurés et les photos « avant-après » ont été placardées sur les murs, afin que la population terrorisée ne sorte plus de chez elle. La liste des atrocités commises s'allonge tous les jours. Elles nous heurtent et nous choquent profondément. La haute-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme a appelé fin septembre à une action urgente pour empêcher que la situation au Myanmar ne se transforme en conflit total. Son bureau a publié un nouveau rapport qui détaille les violations généralisées commises contre le peuple, dont certaines pourraient constituer des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre.

plus rien n'est fait contre le virus qui fait aujourd'hui des ravages terribles. La plupart des hôpitaux civils sont fermés et aucun médicament, vaccin ou oxygène n'est distribué. Puisque les soignants ont été parmi les premiers à entrer en résistance contre le coup d'État, nombre d'entre eux ont été arrêtés ; plusieurs centaines d'autres seraient toujours visés par des mandats d'arrêt. Dans ce contexte, la population continue à se battre pour son droit à la démocratie. Nous ne pouvons pas l'abandonner à son sinistre sort, alors que le pouvoir birman fait brûler des maisons et des villages et piège le terrain avec des mines. De fait, le temps profite aux militaires qui paraissent en position de force et semblent en passe de s'installer pour durer. Ils parient sur un pourrissement de la situation dans le temps long, qui conduirait certains pays à vouloir normaliser leurs relations avec les autorités en place sans pour autant explicitement les cautionner.

en l'état actuel, le Gouvernement d'unité nationale et ses représentants, pour réenclencher un processus de transition démocratique. La France entretient des contacts réguliers avec ce Gouvernement d'unité nationale. Ainsi, la commission des affaires étrangères du Sénat a auditionné le 30 juin dernier plusieurs de ses membres. Parmi les attentes qu'ils ont exprimées devant la commission, celle concernant la nécessité de reconnaître

Vous comprendrez donc le sens de cette proposition de résolution. Pour monter l'attention du Parlement français, un texte quasi identique a d'ailleurs été déposé à l'Assemblée nationale par des collègues députés.

avec les États-Unis et la Chine, comme l'actualité internationale nous le commande. Monsieur le ministre, nous comptons sur vous. La

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en quelques mois, la Birmanie est passée de l'espoir au désespoir. La participation massive des Birmans aux élections de novembre 2020 avait conduit à la victoire de la Ligue nationale pour la démocratie. Ce résultat aurait pu consolider la fenêtre progressiste ouverte en 2015 par quelques généraux réformateurs. Hélas, en février dernier le coup d'État de l'armée birmane est venu plonger le pays dans un chaos que les auteurs de la proposition de résolution ont rappelé : répression, assassinat, détention ou déplacement guettent tous ceux qui contestent le nouveau régime. La situation sécuritaire est en effet dramatique. À travers tout le pays, les forces armées birmanes répriment des manifestations pourtant pacifiques. Alors que les généraux prétendaient seulement vouloir assurer le transfert du pouvoir, ils n'ont fait que déclencher un séisme politique et humanitaire largement condamné sur la scène internationale. Au-delà des atteintes aux droits de l'homme qui nous émeuvent au premier rang, c'est aussi la situation économique qui nous inquiète. Cela a été souligné : l'économie est au point mort. (ONG) et les agences de l'ONU font état de conséquences dramatiques. Le Programme des Nations unies pour le développement constate une aggravation de la pauvreté, et le Programme alimentaire mondial alerte sur la hausse des foyers de malnutrition. Cette crise est un véritable retour en arrière pour les Birmans. Malgré une situation compliquée, malgré les risques, malgré les moyens de la junte, force est de reconnaître le courage de la population, dont une grande partie a entendu l'appel à la désobéissance civile formulée par le Gouvernement d'unité nationale. Entre la dictature et la révolution, le peuple birman a choisi. Il a choisi la liberté, et même les armes à travers la « force de défense populaire ». Dans ces conditions, le soutien de la communauté internationale est indispensable pour appuyer cette quête de liberté. Le groupe du RDSE est donc naturellement favorable à toutes les initiatives dans ce sens. Mais quelles sont les options ? Disons-le, elles ne sont pas nombreuses. Il y a bien le régime de sanctions que la communauté internationale a mis en place depuis mars dernier. Mais nous savons combien les généraux ont imbriqué les intérêts militaires et les intérêts économiques du pays, notamment à travers les fameux conglomérats de l'armée et le Conseil administratif de l'État. Monsieur le ministre, comment cibler les sanctions sans aggraver la situation humanitaire ? Comment également obtenir un soutien plus net des acteurs de la région ? Je pense en particulier à l'Association des nations d'Asie du Sud-Est, dont certains des membres détournent les yeux tandis que d'autres normalisent leurs relations avec la junte. Que penser également de la Chine et de la Russie, qui se sont abstenues lors du vote de la résolution de l'ONU du 18 juin dernier ? Sans avoir souhaité le coup d'État, ces deux puissances autoritaires et décomplexées sont fort logiquement mal à l'aise quand il s'agit d'appuyer le retour à la démocratie à l'extérieur, sans parler de leurs intérêts géostratégiques.

Fidèle à ses valeurs, la France, avec l'appui qu'elle doit rechercher de la part de ses partenaires européens, ne peut qu'apporter son soutien à une représentation qui émane des élections libres de 2020. Mon groupe, je l'ai dit, est favorable à toute démarche qui aiderait le peuple birman à reprendre son destin en main grâce à un gouvernement civil qui, en outre, a donné des gages d'intégration de toutes les minorités ethniques du pays dans un cadre fédéral. Mes chers collègues, le RDSE votera donc la proposition de résolution. Le coup d'État birman constitue une véritable infraction aux conventions internationales. Nous devons notre soutien au peuple birman qui fait preuve d'un grand courage et d'une détermination à retrouver le chemin de la démocratie. J'ajouterai que l'issue de cette crise pourrait également démontrer la capacité de la communauté internationale à maintenir la stabilité dans la zone Asie-Pacifique,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, après les élections de novembre 2020 remportées par la Ligue nationale pour la démocratie, l'armée birmane a pris le pouvoir par la force le 1 février dernier. Depuis cette date, la police et l'armée n'hésitent pas à réprimer par la force toute opposition. En six mois, près de 1 000 civils dont 75 mineurs ont été abattus, des centaines d'entre eux ont disparu et plus de 5 400 personnes sont derrière les barreaux. Malgré cette dureté du régime, la résistance continue de s'organiser courageusement face à la dictature. Il est donc nécessaire d'intensifier les efforts de la communauté internationale pour soutenir les démocrates birmans. Je vais aborder successivement l'action de l'ONU, puis celle de l'Union européenne, et enfin celle de la France. Concernant l'action de l'ONU, non seulement la résolution de l'Assemblée générale adoptée fin juin pour appeler tous les États membres à empêcher l'afflux d'armes vers le pays n'est pas contraignante, mais la Russie et surtout la Chine ont de surcroît bloqué toute résolution ferme au Conseil de sécurité : la ligne de front entre l'autoritarisme- et c'est un euphémisme -dont la Chine est le centre, et l'aspiration démocratique commune à tant de peuples en Asie passe aujourd'hui par les rues de Rangoon, comme elle est passée hier par celles de Hong Kong et de Bangkok. Certes, lors de l'Assemblée générale en cours, la Birmanie- tout comme l'Afghanistan d'ailleurs -a été retirée de la liste des discours, et l'ambassadeur choisi par Aung San Suu Kyi a conservé son siège auprès de l'ONU.

Premièrement, arrêter les flux de fonds vers les militaires birmans, en imposant des sanctions ciblées aux entreprises commerciales de la junte, notamment la, principale source de revenus de l'État birman. Deuxièmement, imposer un embargo international sur les armes. Troisièmement, établir la responsabilité des crimes commis par le biais des tribunaux nationaux ayant recours à la compétence universelle, si le Conseil de sécurité refusait de renvoyer l'affaire devant la Cour Quatrièmement, travailler directement avec la société civile locale et les ONG pour fournir une aide humanitaire. Cinquièmement, enfin, ne pas reconnaître la junte militaire en tant que gouvernement légitime représentant le peuple du Myanmar. On sait que la junte birmane ne changera son comportement que si son moteur économique, et donc financier, est menacé par la communauté internationale. Les mesures à prendre devraient donc inclure non seulement des sanctions ciblées et un embargo international sur les armes, mais surtout des restrictions financières pour réduire les revenus de la junte issus des industries extractives.

peu plus de 20 millions d'euros, et a aussi annoncé des sanctions individuelles contre des responsables du coup d'État ainsi que contre des entités économiques liées à l'armée. Ces mesures visent bien sûr à limiter la capacité de la junte à tirer profit des ressources naturelles du pays. L'Union européenne peut-elle faire plus ? Malgré son poids économique considérable, elle joue hélas un rôle minime sur la scène internationale. Souvent caricaturée comme un géant économique, mais un nain politique, l'Union européenne peine à transformer sa force économique en influence diplomatique,

Pour autant, avec la Birmanie, l'Union européenne a une occasion de plus à saisir pour faire davantage entendre sa voix dans le monde, pour défendre son approche multilatérale jamais démentie, et exprimer sa volonté de faire respecter le droit international.

C'est en réalité une position biaisée, gênée, entravée par la présence de Total dans un conglomérat d'exploitation de gaz, source précieuse de liquidités pour les militaires putschistes. putschistes. En mai dernier, Total a annoncé que les actionnaires d'un gazoduc qu'il exploite en Birmanie allaient cesser de percevoir des versements- parmi eux figure une entreprise liée à l'armée birmane. Le groupe pétrolier a précisé qu'il allait continuer ses opérations en Birmanie, mais qu'il respecterait les sanctions internationales si elles venaient à être prises. Si cette mesure est saluée par les ONG, son impact reste cependant sur le comportement de la junte. C'est donc l'ensemble de ses paiements à la junte que Total doit suspendre. La France doit adopter une approche volontariste et proactive pour atteindre cet objectif. Comment faire ? Une solution

correspondantes sur un compte protégé. Cet argent serait alors conservé jusqu'à ce que la Birmanie ait un gouvernement légitime et démocratiquement élu. En conclusion, malgré les efforts de l'Asean, les sanctions européennes et les condamnations du G7 ou de l'ONU, la crise perdure et la démocratie est confisquée en Birmanie, où le peuple s'enfonce dans la violence et la souffrance. Avec cette résolution, la France appelle à la libération sans condition des prisonniers et à une reconnaissance du Gouvernement d'unité nationale de Birmanie. Pour que la France regagne l'estime des peuples qui attendent beaucoup d'elle, notamment en Asie, ce sont les libertés et les droits de l'homme qu'elle doit défendre

monsieur le ministre, mes chers collègues, en 1962, quatorze ans après son indépendance, un premier coup d'État a stoppé l'élan démocratique en Birmanie. En 2011, brève respiration : la junte laisse en apparence le pouvoir à la société civile.

En dépit de ses efforts, et pour reprendre les mots de l'ambassadeur Christian Lechervy, auditionné par le Sénat le 10 février 2021, « jamais la cohabitation civilo-militaire n'a été harmonieuse durant ces cinq années d'existence Voyant s'approcher le seuil des 75 % de l'Assemblée contrôlés par l'opposition, la junte procède à un coup d'État le 1 février 2021. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont manifesté à Rangoon, à Mandalay et dans plusieurs autres villes. La loi martiale y a été décrétée. Une résistance s'est organisée autour du Gouvernement d'unité nationale, né d'une initiative parlementaire de députés déchus et de plusieurs ethnies minoritaires, avec à sa tête Aung San Suu Kyi et le président de la République Win Myint, toujours emprisonnés. que nous discutons aujourd'hui invite le Gouvernement, premièrement, à travailler avec ses partenaires européens afin d'obtenir une condamnation générale vigoureuse du coup d'État du 1 février 2021 et des violences qui l'ont suivi deuxièmement, à appeler au respect de la démocratie et au rétablissement de la paix ; troisièmement, à reconnaître le Gouvernement d'unité nationale de Birmanie pour l'aider à rétablir la paix. Or, entre le moment du dépôt de cette proposition de résolution et aujourd'hui, de larges changements ont eu lieu, de prendre quelques précautions. D'abord, nous pouvons nous féliciter que la France et ses partenaires européens aient réagi rapidement en appelant à soutenir les actions pacifiques en faveur de la démocratie. Jean-Yves Le Drian a condamné avec la plus grande fermeté ces événements, y compris au Sénat le 3 février dernier. En raison des blocages russes et chinois, aucune déclaration commune n'a pu être arrêtée en février par le Conseil de sécurité des Nations unies. Le 10 mars, il a toutefois fermement condamné les violences. Puis, le 18 juin, l'Assemblée générale a adopté une résolution condamnant le coup d'État. Par ailleurs, les 22 mars, 19 avril et 21 juin, l'Union européenne a imposé des restrictions individuelles aux trente plus hauts responsables et entreprises de la junte, en les interdisant de territoire et en gelant leurs avoirs financiers. Les deux premiers points de la proposition de résolution ont donc déjà trouvé une réponse. Ensuite, le niveau de tensions a augmenté d'un cran : dans ses plus récentes déclarations, le Gouvernement d'union nationale qui était jusqu'alors pacifique appelle désormais à une « guerre défensive », c'est-à-dire à une lutte armée contre les forces de la junte. Cet appel a été critiqué, notamment par le Royaume-Uni, qui a condamné, par un communiqué, « une démarche de nature à éloigner encore davantage l'ouverture de l'indispensable dialogue entre les deux parties Le 30 juin, la commission des affaires étrangères du Sénat a auditionné des membres du Gouvernement et du Parlement birman en exil. Soutenir les actions du Gouvernement d'unité nationale aujourd'hui ne reviendrait-il pas à verser verser de l'huile sur le feu et à cautionner un conflit armé dans lequel nous ne sommes pas engagés directement, alors même qu'il va contribuer à ralentir le processus de stabilisation et à amplifier la crise humanitaire ? Car, enfin, la détresse humaine découlant de cette situation s'est aggravée. Le groupe RDPI tient à réaffirmer tout son soutien à la population birmane, et s'alarme de ces terribles réalités : 25 % de la population et 34 % des enfants

Nous avons conscience que le droit international ne reconnaît que les États, et non les gouvernements, et nous avons vu les limites morales de ce soutien inconditionnel au Gouvernement d'unité nationale. Pour toutes ces raisons, le groupe RDPI opte pour l'abstention, mais laisse chacun de ses membres voter selon leur appréciation personnelle. Néanmoins, monsieur le ministre, plusieurs leviers d'action demeurent utilisables. D'abord, en plus de la pression sur les intérêts financiers de la junte, est-il prévu à moyen terme d'agir sur la préférence tarifaire en retirant le pays du programme « Tout sauf les armes », comme cela a été fait pour le Cambodge ? où en est la revue de l'aide au développement pour éviter son détournement par la junte ? Enfin, quel tournant le dialogue diplomatique avec les autres États membres de la communauté internationale va-t-il prendre, notamment concernant l'embargo sur les armes ? La parole

Quelques années seulement après le début de la transition, l'armée est revenue au pouvoir, et Aung San Suu Kyi est retournée en résidence surveillée. L'armée n'a pas supporté de voir son rôle politique marginalisé par le résultat des élections de novembre 2020, s'emparant du pouvoir par la force, ouvrant le feu sur le peuple qu'elle a pour mission de protéger. Après deux mois de manifestations réprimées à balles réelles, on dénombrait près d'un millier de morts et plusieurs milliers de personnes en détention arbitraire. Le Président de la République a immédiatement condamné ce coup d'État, appelant à mettre un terme à la répression. L'Union européenne s'est insurgée avec la plus grande fermeté contre ce coup d'État militaire. La situation est d'autant plus dramatique que ce putsch intervient dans le contexte de la pandémie. Difficile à gérer en temps de paix, la situation devient catastrophique lorsque l'État est désorganisé. La campagne de test, de et de traitement s'est brutalement arrêtée. Les Nations unies estiment que seulement 40 % des capacités médicales du pays sont encore fonctionnelles. Mauvais augure s'il en est, la junte a commencé récemment la construction de dix crématoriums. Cette prise de pouvoir est une catastrophe pour la population et sa santé, mais aussi pour son économie. Elle déstabilise une économie déjà fragile. Près de la moitié des habitants sont susceptibles de se trouver sous le seuil de pauvreté d'après les Nations unies. La situation nécessiterait l'envoi d'aide humanitaire, mais, même si cette dernière parvenait jusqu'au territoire birman, rien ne garantit qu'elle bénéficierait effectivement au peuple. Cette situation constitue également un défi à la stabilité de la région. La Chine possède de nombreux intérêts en Birmanie, et son influence y est considérable. Pékin entretenait de bonnes relations avec le gouvernement précédent, ce qui ne l'a pas empêché de qualifier le coup d'État de simple « remaniement ministériel ». Le tracé des nouvelles routes de la soie emprunte le territoire birman. C'est dire à quel point la stabilité de ce pays, mais non la ce n'est pas Pascal Allizard qui dira le contraire ! La junte précédente a pu faire face aux sanctions occidentales principalement grâce au commerce avec son grand voisin. Tant qu'elle pourra assurer une relative stabilité dans le pays, la junte actuelle ne sera pas inquiétée par la Chine. La légitimité de la junte reste cependant très contestée, tout d'abord démocratiquement par le Gouvernement d'unité nationale, constitué de parlementaires élus lors des dernières élections, mais forcés à l'exil. Elle l'est également par les armes, au travers d'une lutte engagée par des mouvements de guérilla. Même ceux qui avaient conclu un cessez-le-feu ont repris le combat dès le mois de mars ; certains se sont emparés de bases militaires et de commissariats de police. Ces mouvements sont structurés autour de milices ethniques. La Birmanie compte, à côté de l'ethnie majoritaire birmane, plus d'une centaine de minorités, dont l'incorporation dans une seule et même nation reste inachevée. La voie démocratique permettait à chacun de s'exprimer et d'espérer peser sur la politique du pays. Le retour de la junte, c'est le retour de la force, le retour des affrontements. Face à cette triple urgence- humanitaire, économique et démocratique nous ne sommes pas démunis : sans avoir le poids de la Chine, nous pouvons et nous devons appeler à la reconnaissance du gouvernement d'unité nationale. Ce gouvernement inclusif est en effet le plus à même de garantir la stabilité d'un pays marqué par les conflits ethniques, que seule la transition démocratique avait permis d'apaiser. Des sanctions économiques ont été prises ; d'autres doivent venir les renforcer. Nous devons toutefois continuer de nous assurer qu'elles pénalisent les responsables de la junte en épargnant le peuple. Le groupe Les Indépendants, qui compte des signataires de la proposition de résolution, est convaincu que la reconnaissance du gouvernement d'unité nationale est une étape incontournable dans la résolution de la crise birmane. Nous voterons donc en faveur de cet excellent texte. La

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

Je félicite donc mon collègue pour ses qualités de persuasion ayant abouti à ce que le groupe Les Républicains accepte le dépôt de cette proposition de résolution et son inscription à notre ordre du jour. Déposer et débattre d'une proposition de résolution relative à la Birmanie est un exercice de diplomatie parlementaire quelque peu difficile, mais c'était indispensable au regard de la situation dramatique dans ce pays, sur laquelle je ne reviendrai pas, ayant déjà beaucoup parlé et écrit à ce sujet.

qu'il fallait absolument avoir une approche globale de la situation, incluant tous les acteurs susceptibles d'oeuvrer pour le rétablissement de la paix. La toute première des priorités est, bien sûr, l'arrêt des exactions à l'encontre de la population. En juin dernier, mon homologue de l'Assemblée nationale, Alain David, et moi-même avons publié une tribune dans le journal, dans laquelle nous demandions déjà la reconnaissance du gouvernement d'unité nationale et l'affectation des dividendes de Total et du secteur gazier à un compte bloqué.

Pour moi, l'examen de cette proposition de résolution constitue donc autant un appel renouvelé à notre diplomatie que l'occasion d'un point d'étape

Une crise en chassant vite une autre, je crains que les priorités dans les agendas diplomatiques ne divergent largement ... Pouvez-vous également dresser un bilan du troisième train de sanctions, décidé avant l'été Ces sanctions sont indispensables, mais, aujourd'hui, elles semblent nettement insuffisantes pour arrêter l'effusion de sang. Elles affectent durement la population civile et deviennent parfois contre-productives. Nous ne pouvons nous en contenter. En 2007, déjà, j'interrogeais une secrétaire d'État chargée des droits de l'homme sur les revenus de la junte et leurs dépôts dans des places fiscales hors d'atteinte. Hélas, peu a été fait depuis Par ailleurs, je le disais en mars dernier, rien n'évoluera sans une réponse régionale, et la neutralité affichée des pays de l'Asean ne saurait être un prétexte à l'inaction.

compte. Mon avant-dernier point concerne notre action d'urgence, notamment humanitaire. Alors que le Parlement a adopté, en juillet 2021, une loi relative à la politique d'aide au développement- engageant une réorganisation entre les opérateurs, je souhaite connaître les modalités d'action de l'Agence française de développement (AFD) dans le pays et le bilan à long terme des investissements en faveur du développement, si possible avant même la constitution de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement. Il nous faut absolument une mobilisation plus large, économique, bien sûr, mais aussi humanitaire et culturelle. Avant de conclure, je souhaite aborder la situation des responsables politiques. Depuis des années, j'ai ce dossier à coeur et la remise du prix Nobel de la paix à Aung San Suu Kyi restera pour moi un moment d'immense espoir. assignée à résidence et réduite au silence, en attendant son procès pour des motifs fallacieux, qui vont de la corruption à l'importation de talkies-walkies, en passant par le trouble à l'ordre public et le non-respect du protocole sanitaire. Les inquiétudes sur son avenir sont très fortes

À travers elle, je pense également à la relève politique de ce pays. Il importera que, par différents leviers, la France maintienne ses relations et ses actions dans ce pays, afin que la Birmanie ne sombre pas définitivement dans les ténèbres. Nous ne pouvons pas abandonner ce pays. Le peuple birman, si assoiffé de démocratie, si courageux, compte sur nous. Il se bat seul et son courage force l'admiration. Pour enrayer cette guerre civile, qui est déjà enclenchée et ne cesse de s'amplifier, il est indispensable que les Nations unies établissent un embargo sur les armes lourdes, fournies essentiellement par la Russie et par la Chine, que soit renforcé le dialogue avec les EAO (), les groupements ethniques armés, et avec le CDM, le mouvement populaire de désobéissance civile, et, bien entendu, que soit reconnu le gouvernement d'unité nationale. Ce serait pour la Birmanie un immense espoir, de nature à décourager un peu plus l'armée, cette sinistre, qui semble aujourd'hui tétanisée face aux désertions aux attaques de ces Birmans, si courageux et prêts à sacrifier leur vie pour leur liberté. Je vous le disais ici même, en mars dernier, la France a une responsabilité historique : elle se doit d'encourager le valeureux peuple birman en lutte contre une dictature mafieuse elle se doit de montrer au monde qu'elle reste fidèle à ses valeurs de liberté et de droits de l'homme, en entraînant les autres pays à faire de même. En réponse à cela, vous nous aviez parlé, monsieur le ministre, de la détermination de la France à trouver une solution. Vous avez déjà bien agi.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de résolution d'initiative transpartisane dont nous débattons aujourd'hui doit faire l'objet d'un soutien unanime de la Haute Assemblée. Depuis le coup d'État du 1 février dernier, le peuple birman, dans toute sa diversité, a subi une répression d'une violence inouïe. Des millions de personnes sont descendues dans les rues pour s'opposer à la prise de pouvoir de la junte, malgré les menaces de l'armée. Le résultat, huit mois plus tard, est dramatique plus d'un millier de personnes sont déjà mortes sous le feu de l'armée birmane et, au mois de juillet 2021, plus de 250 000 personnes avaient été déplacées. La Birmanie compte ainsi presque 700 000 déplacés internes aujourd'hui, alors qu'elle est déjà minée par les conflits interethniques et par les ravages de la pandémie. Pour compléter ce sinistre tableau, les ONG font état d'arrestations arbitraires par la junte, de disparitions forcées, d'actes de torture et de viols. Ces actes pourraient constituer, au regard du droit international, des crimes contre l'humanité. C'est ce régime brutal et méprisant le droit international qui tentait d'obtenir, encore le mois dernier, un siège à l'Assemblée générale des Nations unies. Cela lui a été refusé, grâce à un accord durement négocié avec la Chine. C'est une bien maigre victoire, car, si la junte est en manque de légitimité internationale aujourd'hui, cela ne l'empêchera pas de se maintenir au pouvoir par la violence. Certes, son autorité est contestée sur des pans entiers du territoire, mais les groupes armés locaux qui se sont formés pour la combattre ne constituent pas un front uni et n'ont pas les moyens de reconquérir le pays. Ne nous laissons pas tromper par les apparences de gouvernement civil dont la junte essaie de se parer ni par ses promesses d'élections d'ici à 2023. Ce pouvoir tyrannique n'offre aucune garantie de stabilité à moyen terme ; il offre plutôt la promesse d'un conflit interne, dont les civils seront les premières victimes. Mes chers collègues, nous ne pouvons pas être optimistes. Les perspectives de retour à la paix semblent lointaines. En effet, le 7 septembre dernier, le président intérimaire du gouvernement d'unité nationale appelait à un soulèvement populaire contre l'armée birmane. Comment pourrait-il en être autrement ? Le gouvernement d'unité nationale représente tout simplement la seule perspective d'un retour à l'État de droit pour le peuple birman. Formé au mois d'avril par le Comité représentant l'Assemblée de l'Union, comité issu des élections de novembre 2020, ce gouvernement est porteur d'une légitimité politique indéniable. Au-delà de cette légitimité tirée des urnes, nous tenons à saluer sa diversité ethnique ; la représentation des minorités et le dialogue interethnique seront une condition pour présenter une solution de substitution crédible à la junte et construire une paix durable dans cette société si fracturée. Nous nous en réjouissons d'autant plus que cela constitue une amélioration notable par rapport au gouvernement de Mme Aung San Suu Kyi, qui, rappelons-le, avait défendu la persécution de la persécution de la population rohingya. À ce jour, ce gouvernement d'unité nationale a démontré à maintes reprises sa volonté et sa capacité de participer aux discussions multilatérales dans les instances internationales. Notre commission des affaires étrangères a même rencontré à distance certains de ses membres. Néanmoins, ce gouvernement a aussi cruellement besoin du soutien de la communauté internationale. Nous avons, certes, condamné la junte à de multiples reprises et à de nombreuses tribunes, et nous l'avons soumise, avec l'Union européenne, à des sanctions économiques. l'opposition à un régime sur lequel nous avons peu de prises et le soutien informel à ce gouvernement d'unité nationale fantôme ne sont plus à la hauteur de la situation. C'est pourquoi le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires votera évidemment pour la présente proposition de résolution. La France doit travailler avec ses partenaires européens pour appeler à une réaction internationale plus forte contre le coup d'État et contre les violences qui l'ont suivi. Elle doit également demander la libération des prisonniers politiques et la fin de l'état d'urgence. Enfin, et surtout, nous avons le devoir de soutenir un gouvernement qui qui a démontré son attachement aux principes démocratiques, à la représentativité de la mosaïque ethnique qui compose la Birmanie et à un dialogue ouvert avec la communauté internationale. Ce sont non seulement les Birmanes et les Birmans que nous défendons en votant pour ce texte, mais également nos valeurs. Pour conclure, j'ajoute que nombreux sont les pays à travers le monde, notamment en Afrique, dans lesquels la France et l'Union européenne devraient soutenir les transitions démocratiques, sans faire le tri en fonction de leurs intérêts militaires et économiques.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis le 1 février dernier, la Birmanie est, une nouvelle fois, dans une situation de chaos. Ce quatrième coup d'État en à peine soixante-cinq ans et la répression que subissent les opposants ont déjà fait plus d'un millier de victimes civiles et plus de quatre mille prisonniers. En parallèle, écoles, hôpitaux et postes de police ont été vidés, la junte militaire décidant de purger les fonctionnaires qui refusaient cette prise de pouvoir illégitime. Quelque 300 000 travailleurs ont été licenciés de façon arbitraire et 25 millions de personnes vivent en situation de pauvreté. Face à cette situation, que faire ? En premier lieu, il me semble essentiel que nous arrivions à une condamnation la plus large possible du coup d'État. C'est ce qui est proposé au travers de cette proposition de résolution, que notre groupe votera.

de sécurité du 4 février allait dans le bon sens, en appelant à l'abandon des violences, au maintien des institutions démocratiques et au respect des libertés fondamentales, elle ne suffisait malheureusement pas. Il aura ainsi fallu attendre le 18 juin pour que les Nations unies condamnent officiellement le coup d'État. De la même manière, l'Union européenne a imposé des sanctions économiques, mais seront-elles suffisantes ? Nous pouvons en effet nous interroger sur la pertinence de la décision consistant à ne pas intégrer certains secteurs essentiels dans le champ des sanctions, tout comme nous devons garder en mémoire la stratégie de la junte, dans les années 1990 et 2000, qui avait creusé les immenses besoins de la population civile. Cette stratégie était d'autant plus cynique que, pour reprendre les termes du chercheur David Camroux, « en 1939, la Birmanie était le plus grand

En deuxième lieu, tous les moyens doivent être mis en oeuvre pour éviter de soutenir, même indirectement, la junte militaire. Ce n'est qu'un premier pas, mais la résolution du 18 juin dernier appelle les Nations unies à empêcher l'afflux d'armes en Birmanie. Espérons que cela se révèle plus efficace que le précédent appel concernant la Libye Surtout, je m'interroge sur le rôle joué par certains grands groupes, notamment états-uniens et français. Si l'enquête parue dans en mai dernier était vraie, ne serait-ce que partiellement, nous serions face à un véritable scandale. Ainsi, le géant pétrolier français, qui exploite depuis 1998 le gisement gazier de Yadana, serait au coeur d'un système grâce auquel des centaines de millions de dollars seraient détournés

La décision de Total, prise sous la pression de nombreuses ONG, de suspendre ses versements aux actionnaires de l'entreprise birmane n'est qu'une micro-réponse à un gigantesque problème.

En troisième et dernier lieu, il est d'ores et déjà nécessaire de penser à l'avenir. On le voit bien, malgré ce qui ressemblait à un accord des deux grandes forces politiques birmanes en faveur de la libéralisation du pays, cette dernière restait fragile. La Birmanie, avant même le 1 février 2021, était un pays fortement divisé et en proie aux conflits internes, non seulement politiquement, comme je l'évoquais, mais aussi entre ses différents groupes de population. Nous devons espérer un retour des instances démocratiques légitimement élues, mais ce simple retour ne saurait suffire. Malgré le dialogue interethnique engagé au printemps 2016, on ne peut pas effacer des décennies de tensions entre les différentes communautés. Les massacres et la déportation de presque 700 000 Rohingyas,

La Birmanie, et en premier lieu certaines de ses minorités, paie encore aujourd'hui le tribut de décennies de stratégie cynique des Britanniques, lorsque ceux-ci occupaient le pays. La France devra soutenir dès que possible, entre autres initiatives, celle de la procureure de la Cour pénale internationale destinée à établir clairement les responsabilités dans les exactions de 2017. Un dialogue interethnique, sous l'égide de l'ONU, pourrait s'avérer une piste sérieuse pour résoudre ce conflit. Toutefois, tout cela ne peut être que corrélé à un retour des instances légitimement élues en novembre 2020 et aujourd'hui condamnées au silence ou à la clandestinité. La

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite tout d'abord remercier notre collègue Pascal Allizard, qui a pris l'initiative de déposer cette proposition de résolution permettant aujourd'hui de nous exprimer sur la situation dramatique à laquelle est confrontée la Birmanie. Ce texte, que nous avons été nombreux à cosigner, vise à rappeler au gouvernement français la nécessité de reconnaître le gouvernement d'unité nationale de Birmanie, dont la constitution a été annoncée le 16 avril 2021, et de lui apporter notre soutien dans ses actions de rétablissement de la paix et de la démocratie. Cet engagement, dans des conditions difficiles, de toutes les oppositions au pouvoir dictatorial, jusque-là divisées, constitue un immense espoir. Pour la première fois dans l'histoire du pays, chacune des principales ethnies y est représentée. Depuis l'arrestation, le 1 février dernier, du président de la république, Win Myint, de sa conseillère, Aung San Suu Kyi, et de centaines d'élus, militants ou personnalités politiques défavorables au régime militaire, la junte birmane a repris le pouvoir par la violence, au mépris de toutes les règles gouvernementales qui devraient pourtant être applicables au pays. Paris a condamné fermement cette remise en cause du processus démocratique engagé depuis une dizaine d'années et a appelé au strict respect des résultats des élections du 8 novembre 2020, largement gagnées par la Ligue nationale pour la démocratie. L'action du G7, la troisième série de sanctions prise par l'Union européenne au mois de juin et la pluie de condamnations internationales n'ont pas suffi à rétablir le calme ou à laisser entrevoir une sortie de crise. En mars et avril derniers, de nombreux manifestants birmans se sont opposés vivement à ce coup d'État, mais le soulèvement citoyen s'est tari, car l'armée, tirant à balles réelles, a provoqué des centaines de morts.

L'économie est exsangue ; le système de soins, le système éducatif et tous les services de base sont de plus en plus défaillants. La violence et les tueries se poursuivent de manière incessante. Les 54 millions d'habitants de la Birmanie font face à des crimes odieux, à la mort et à la destruction. En outre, le Programme alimentaire mondial estime que plus de 6,4 millions de Birmans sont exposés à un risque de famine d'ici à la fin du mois d'octobre. Enfin, nous ne pouvons passer sous silence la vague épidémique de covid-19 qui s'est abattue sur le pays en quelques mois. Avant le coup d'État, la Birmanie avait connu un confinement long permettant de protéger la population. Une campagne de vaccination avait même été lancée en début d'année. Depuis février, plus rien n'est fait ; la gestion de la pandémie par l'armée est désastreuse et le virus tue massivement. Lors de l'audition, par notre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, le 30 juin dernier, des membres du gouvernement d'union nationale et du parlement birman en exil, la question de l'aide humanitaire est apparue primordiale. Les difficultés d'acheminement de cette aide et le risque que ces moyens tombent aux mains de la junte empêchent toute intervention. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire si un plan d'action humanitaire est aujourd'hui envisageable ? Un processus coordonné avec d'autres membres de l'Union européenne peut-il voir le jour ? Plus inquiétant encore est le véritable tournant qui est en train de se dessiner, à la suite de la déclaration du président par intérim du gouvernement d'unité nationale appelant à un soulèvement armé contre les militaires dans tout le pays. Cette prise de parole laisse entrevoir le spectre d'une guerre civile. Aujourd'hui, les militaires ne recueillent absolument pas le soutien du peuple, mais les opposants ne disposent pas des moyens sur le terrain pour dominer. L'importance d'une mobilisation internationale pour stopper cette escalade de la violence est capitale. Pourtant, la dernière Assemblée générale de l'ONU n'a pas permis d'avancée majeure : l'ambassadeur birman nommé par le gouvernement civil renversé a conservé son siège auprès de l'ONU, soutenu par la communauté internationale, mais n'a pas pu s'exprimer. La junte, de son côté, a nommé un ex-militaire pour le remplacer, mais cette décision n'est pas entérinée par l'ONU à ce jour ; ce devrait durer au moins jusqu'au mois de novembre. Les discussions à l'échelon régional ne sont guère plus encourageantes. La feuille de route en cinq points, adoptée lors du sommet de l'Asean du 24 avril dernier et visant à mettre un terme aux violences et à trouver une sortie de crise négociée, n'est absolument pas respectée par la junte. Le fait que les pays qui composent cette association soient gouvernés par des régimes politiques très différents, pas tous démocratiques, ne simplifie rien. La règle du consensus préalable à toute décision paralyse les prises de position claires en faveur du gouvernement d'union nationale birman. Alors que les multiples efforts diplomatiques ont montré certaines limites, d'autres actions doivent être envisagées. L'affaiblissement des moyens financiers de la junte constitue certainement le meilleur moyen pour stopper la barbarie et pour entamer un dialogue de sortie de crise. Les sanctions économiques prises par les pays étrangers touchent les dirigeants militaires par le blocage de leurs avoirs personnels. Cependant, la Chine, dont les intérêts économiques et stratégiques directs en Birmanie sont importants, dispose d'une influence incontestable dans l'évolution à venir de ce conflit. Même si la position de Pékin reste floue, son soutien penche davantage vers le gouvernement militaire. En achetant notamment le teck, le jade et les métaux rares, la Chine lui apporte des devises. On peut également s'interroger sur le positionnement de groupes pétroliers qui continuent de verser des sommes énormes aux putschistes, permettant de ce fait à ces derniers de rémunérer les militaires et les policiers. Total s'était engagé, avant l'été, à verser en compensation le montant des impôts et des taxes aux organisations humanitaires. Les mois passent, mais rien n'est fait en ce sens. Il est important de rappeler que, actuellement, l'apport financier du secteur des hydrocarbures à un pouvoir illégitime responsable des pires exactions demeure un réel problème à résoudre rapidement. Les acteurs économiques doivent, eux aussi, réfléchir aux moyens de priver l'armée birmane de revenus. Pour conclure, cette proposition de résolution, au-delà de l'envoi d'un signal politique fort de soutien à la Birmanie, doit permettre d'encourager notre exécutif et, plus largement, nos partenaires diplomatiques à se mobiliser. À l'heure où de grandes ethnies et même, ces derniers jours, l'Arakan- aussi connu sous le nom de Rakhine -ont fait acte d'allégeance au gouvernement d'union nationale, leurs armées progressent dans cinq grandes zones de rébellion et contrôlent de plus en plus de territoires. L'espoir subsiste et nous devons l'accompagner. La parole est à M.

mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de me donner la possibilité d'échanger avec vous sur la situation en Birmanie à la suite du coup d'État du 1 février 2021 en discutant

Votre proposition de résolution témoigne de l'intérêt constant de la société française et de ses représentants pour cette crise. Elle constitue une expression de notre solidarité avec le peuple birman, dans ces instants d'une difficulté particulière. La France est profondément préoccupée par la dégradation de la situation politique et des droits de l'homme en Birmanie depuis le coup d'État, le coup d'État, qui fut une négation de la volonté que le peuple birman avait exprimée lors des élections générales du 8 novembre 2020, du 8 novembre 2020, une grave atteinte à l'État de droit et aux principes démocratiques, que la France a condamnée avec la plus grande fermeté, et ce à de nombreuses occasions. Pour ces raisons, comme la France l'a déjà exprimé à plusieurs reprises, nous ne reconnaissons aucune légitimité au régime issu du coup d'État. Cette position est partagée par nos partenaires européens. Par ailleurs, nous sommes très préoccupés par la dégradation de la situation humanitaire en Birmanie. La répression menée par les forces de sécurité cible en particulier les défenseurs des droits, les journalistes, les représentants des organisations de la société civile et le personnel médical. En particulier, les exactions menées contre le personnel médical, qui a largement rejoint le mouvement de désobéissance civile après le 1 février, affaiblissent la capacité du pays à répondre à la deuxième vague de l'épidémie de covid-19, qui sévit depuis l'été 2021 ; certains d'entre vous y ont fait référence.

Elle fait face à plusieurs accusations arbitraires : corruption ; violation des lois relatives à l'état d'urgence sanitaire et au confinement ; importation illégale de matériel réglementé. Les audiences de son procès ont eu lieu deux fois par semaine en juin, puis une décision de report a été prise à la mi-juillet en raison de la situation épidémique. Celles-ci ont repris en septembre. La conseillère d'État a d'ailleurs indiqué avoir été vaccinée, alors qu'elle était en résidence surveillée. La France s'est mobilisée dès le premier jour pour répondre à cette crise. Nous avons été particulièrement actifs pour pousser la communauté internationale à prendre une position claire et unie sur la situation en Birmanie, une position fondée sur le respect et la protection des droits de l'homme. La résolution adoptée à la quasi-unanimité par l'Assemblée générale des Nations unies, le 18 juin dernier, témoigne du fait que l'attention portée par la communauté internationale à la Birmanie n'a en rien fléchi depuis six mois. Cette résolution va encore plus loin que les déclarations du Conseil de sécurité : elle appelle tous les États qui ne l'auraient pas déjà fait à imposer un embargo sur les livraisons d'armes vers la Birmanie.

Par ailleurs, la France a joué un rôle moteur dans la réponse européenne. Les deux premiers volets de sanctions, chère Joëlle, adoptés en mars et avril derniers, ciblent d'ores et déjà vingt les deux principaux conglomérats militaires- la (MEC) et la (MEHL) -et leurs trente-quatre filiales détenues à plus de 50 % dans des secteurs aussi diversifiés de l'économie birmane que les pierres précieuses, la finance ou le commerce. Le Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne a adopté, le 21 juin, un troisième volet de sanctions qui cible huit nouveaux individus liés au coup d'État et quatre entités économiques. Sont notamment visées des entreprises publiques dans le secteur du bois et des pierres précieuses, ainsi que la principale organisation gérant les actifs des vétérans des forces armées. Comme vous le voyez, nous sommes déterminés, avec nos partenaires européens, à maintenir la pression sur le régime issu du coup d'État. qui concerne les sanctions commerciales, aucune piste n'est écartée, y compris la suspension du régime européen « Tout sauf les armes », chère Nicole Duranton. Ces sanctions doivent respecter deux principes : frapper la junte militaire et éviter de pénaliser la population civile et les emplois induits par les exportations vers l'Union européenne. Au-delà des sanctions, nous avons suspendu tout soutien budgétaire aux programmes gouvernementaux. Nous n'écartons aucune option, y compris en matière de préférence commerciale. commerciale. Nous prenons acte des décisions de Total. Comme je l'indiquais, notre position est sans ambiguïté : frapper les intérêts économiques des forces de sécurité birmanes tout en préservant la population civile.

L'entreprise a réaffirmé à cette occasion, comme l'ont rappelé certains d'entre vous, qu'elle respectera toute décision qui pourrait être prise par les organisations internationales ou nationales compétentes, y compris les sanctions imposées par les autorités européennes et américaines.

: pas de nouveaux transferts financiers ; pas de nouvel accord ; pas de contact de haut niveau. En revanche, nous avons poursuivi les projets d'appui à la société civile.

que la situation sanitaire se dégrade, la France continuera d'apporter son soutien à la société civile et maintiendra son aide humanitaire. En ce qui concerne la reconnaissance du gouvernement d'unité nationale, la position de la France est claire et constante : elle ne reconnaît que les États, et non les gouvernements. Cette position est d'ailleurs partagée par l'ensemble de nos partenaires européens. À ce jour, aucun État n'a reconnu le gouvernement d'unité nationale, malgré les efforts déployés par ses membres. Cela étant, nous n'avons ménagé aucun effort pour valoriser le travail de cette structure, qui émane du Comité représentant l'Assemblée de l'Union (CRPH), dont les membres ont été démocratiquement élus. Nous nous efforçons également de lui donner une tribune dans les enceintes multilatérales. Ainsi, Susanna Hla Hla Soe, ministre des femmes, de la jeunesse et de l'enfance, a pu s'exprimer lors de la séance publique du Conseil de sécurité des Nations unies, le 29 juillet dernier, pendant la présidence française. La France souhaite que le gouvernement d'unité nationale et le CRPH fassent partie du futur processus politique de dialogue, qui permettra une sortie de crise. Nous ne ménageons pas nos efforts pour l'affirmer publiquement ni pour amener l'Union européenne à le faire. Je vous renvoie ainsi à la déclaration du 30 avril Haut Représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, sur les résultats de la réunion des dirigeants de l'Asean. Aux Nations unies, la représentation de la Birmanie fait aussi l'objet de toute notre attention. La France n'est pas représentée à la commission de vérification des pouvoirs pour la session de cette année, mais sa position est claire.

à la junte. Si nous partageons la plupart des principes et objectifs de la proposition de résolution, la position de la France, je le répète, demeure constante : elle ne reconnaît pas les gouvernements, mais seulement les États. Pour ces raisons, je m'en remets à la sagesse du Sénat.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en présentant voilà un an son pacte sur les migrations et l'asile, la Commission proposait à l'Europe de prendre un « nouveau départ », à la faveur duquel elle pourrait enfin tourner la page tourner la page : celle des carences profondes du système de gestion des frontières extérieures et de l'asile, révélées par la crise de 2015, et celle de la division, qui a empoisonné les relations entre États membres et conduit à l'enlisement du précédent paquet Asile. Le groupe Les Républicains fait naturellement sienne cette ambition de s'attaquer aux principaux maux ayant plongé l'Europe dans un tragique état de fragilité face aux phénomènes migratoires. Dans un contexte où les flux migratoires vont encore s'accroître en raison du changement climatique ou de l'explosion démographique de l'Afrique, l'enjeu est évidemment immense. Il est tout d'abord intérieur, car il engage la crédibilité même du projet européen vis-à-vis de nos concitoyens, qui gardent encore en mémoire l'incapacité de l'Union à faire face efficacement à la crise des réfugiés. Souvenons-nous qu'alors, ce sont les fondations mêmes de l'espace Schengen qui vacillèrent, menaçant d'emporter avec elles le principe de libre circulation et installant la question migratoire comme une question existentielle pour l'Union européenne. Mais l'enjeu est également extérieur, certains de nos voisins n'hésitant plus à exploiter nos failles et à transformer les migrations en arme géopolitique. La Turquie fut la première à en user, tant pour s'assurer de la retenue des Européens face à sa politique expansionniste que pour en tirer de substantiels revenus- 6 milliards d'euros ont ainsi été versés depuis 2016 et 3,5 milliards d'euros devraient suivre prochainement. Depuis, ce chantage migratoire a fait des émules : c'est désormais au Maroc et à la Biélorussie de s'essayer à la même méthode pour obtenir de l'Union ou des États membres une inflexion de leur politique étrangère. Face à ces défis, la réponse européenne doit bien évidemment se déployer sur de multiples fronts, mais elle doit avant tout envoyer un message clair et affirmer ce principe cardinal : nul ne doit pouvoir entrer ou s'installer sur le sol européen sans y avoir été au préalable légalement autorisé. La constitution d'un système européen robuste, en mesure de faire respecter ce principe, quelles que soient les circonstances, est donc la première des priorités. Les États membres qui sont, et qui doivent rester les seuls maîtres de leur politique migratoire et de leurs frontières en seront les principales chevilles ouvrières. Comme toujours en matière européenne, c'est de leur implication que dépendra la réussite, ou l'échec, de la politique menée. À ce titre, le pacte prévoit un renforcement du cadre de gouvernance afin de mieux identifier les éventuelles lacunes. Si nécessaire soit-elle, cette approche sera-t-elle pour autant suffisante ? On peut en effet s'interroger, dans la mesure où, en l'absence de régime contraignant, le système proposé ne reposera que sur la pression des pairs et sur l'engagement de la Commission à recourir aux procédures d'infraction à l'encontre des États qui ne rempliraient pas leurs obligations légales. Bien évidemment, l'Europe ne peut se contenter de surveiller ou de sanctionner les États membres. Elle doit avant tout être pour eux un levier leur permettant de retrouver des marges de manoeuvre, tant au niveau des moyens mis à leur disposition que des procédures applicables en matière d'asile et de retour. Des avancées ont d'ores et déjà été enregistrées en la matière. Je pense, en premier lieu, à la création prochaine de l'agence européenne pour l'asile, ainsi qu'à celle, fin 2016, du corps européen de garde-côtes et garde-frontières, dont la montée en puissance doit s'accélérer. Je pense également à la création de nouveaux systèmes de contrôle aux frontières, à l'interconnexion des bases de données numériques ou encore au doublement, dans le cadre financier pluriannuel, des fonds dédiés à la gestion des migrations et des frontières. En ce qui concerne les procédures, les propositions du pacte me semblent aller plutôt dans le bon sens. Ainsi, les nouvelles procédures de filtrage et d'asile à la frontière, couplées à l'élargissement de la base de données Eurodac et aux précédentes propositions de révision des directives Accueil, Qualification et Procédures, devraient permettre aux États membres d'agir plus efficacement. En n'étant pas tenus d'autoriser l'entrée sur leur territoire et en recourant plus aisément au placement en rétention, ces derniers pourront opérer un contrôle plus strict des demandes d'asile et des mouvements secondaires. Ils pourront également distinguer plus rapidement les personnes pouvant légitimement prétendre à la protection internationale de celles qui ont vocation à être reconduites dans leur pays d'origine. Cette nouvelle orientation est d'autant plus essentielle que seules 39 % des demandes d'asile formulées dans l'Union européenne en 2018 avaient reçu une décision positive en première instance. Toutefois, le nouveau règlement sur la gestion de l'asile et des migrations, proposé en remplacement du très décrié règlement de Dublin, appelle à davantage de circonspection. La proposition a le mérite d'abandonner définitivement l'idée des quotas de migrants, qui a contribué à tendre à l'extrême les relations entre États membres et qui, de ce fait, était vouée à l'échec.

Cette grande complexité est sans doute le prix à payer pour tenter de concilier des points de vue diamétralement opposés, mais elle risque de nuire à l'efficacité et à la lisibilité de l'ensemble. Enfin, soulignons que la crédibilité du dispositif reposera en grande partie sur l'amélioration de la politique de retour. À ce jour, les chiffres sont catastrophiques : seuls 29 % des personnes qui reçoivent chaque année l'ordre de quitter l'Union européenne regagnent effectivement leur pays,

il est consternant que le poste de coordinateur de l'Union européenne pour les retours, annoncé lors de la présentation du pacte, n'ait toujours pas été pourvu à ce jour. Le renforcement de nos procédures et de nos moyens internes, pour s'assurer de la rapidité et de la bonne exécution des décisions de justice, est donc fondamental. Cependant, une fermeté accrue dans le volet extérieur de cette politique de retour est tout aussi indispensable. La révision du code des visas, adoptée en 2019, qui propose de durcir ou, au contraire, d'assouplir l'octroi de visas en fonction de l'effectivité des réadmissions, montre la voie à suivre. La logique mérite aujourd'hui d'être étendue à d'autres leviers, tels que les accords commerciaux et les politiques d'aide au développement, pour s'assurer une bonne coopération des pays tiers en matière de prévention des migrations ou de réadmission des migrants irréguliers. irréguliers. Madame le ministre, mes chers collègues, après cinq ans de négociations infructueuses et de psychodrames, l'Europe ne peut plus se permettre, sur un sujet aussi primordial pour nos concitoyens, le luxe de la désunion, de l'attentisme et de l'inefficacité. Lors de la précédente présidence française du Conseil, en 2008, Nicolas Sarkozy avait réussi, malgré les obstacles, à convaincre ses partenaires d'adopter un texte déjà intitulé « pacte sur l'immigration et Ce pacte a aujourd'hui besoin d'être réformé pour faire face à l'amplification du problème migratoire. Souhaitons que la prochaine présidence française de l'Union se montre à la hauteur de l'enjeu. La parole

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais tout d'abord remercier le groupe Les Républicains d'avoir souhaité provoquer ce débat devant la Haute Assemblée. Il est pour nous l'occasion d'échanger et de revenir sur la détermination du Gouvernement à agir pour renforcer l'espace de liberté et de sécurité que doit constituer l'Union européenne. Chacun le constate, la réponse à apporter aux flux migratoires récents, actuels et à venir, est une préoccupation majeure de nos concitoyens. Notre politique européenne commune en matière d'asile et d'immigration doit être revue en profondeur

2016. Comment faire ? La France appelle depuis longtemps de ses voeux une réforme ambitieuse pour deux raisons principales. D'une part, parce que notre espace de libre circulation- une des conquêtes les plus précieuses de la construction européenne -appelle des règles communes : on ne peut avoir une frontière extérieure commune, un espace sans frontières intérieures et se satisfaire de la disparité actuelle des pratiques des États membres. D'autre part, parce que notre environnement est de plus en plus difficile. Les migrations internationales apparaissent comme un phénomène incontournable qui doit être régulé. Nous devons aussi avoir à l'esprit que les flux migratoires alimentent des filières criminelles très prospères qui se nourrissent de la misère humaine. Enfin, ces flux sont désormais souvent utilisés contre nous par certains États, avec beaucoup de cynisme- nous l'avons vu l'été dernier avec la Biélorussie. Ne croyons pas, cependant, que l'Europe soit restée passive depuis 2015 : je pense, en particulier, au règlement Frontex de 2019, qui nous a permis de doter l'agence de moyens considérables. Nous en déjà débattu ici même. C'est d'ailleurs pour faire face à ces défis que la Commission européenne a proposé, le 23 septembre 2020, un pacte européen sur les migrations et l'asile. et l'asile. Le Gouvernement est convaincu que cette proposition ambitieuse contient les outils qui vont nous permettre de mettre en place une politique migratoire européenne ambitieuse et cohérente. Par rapport au paquet Asile de 2016, dont la négociation avait fini par s'enliser, je relève une différence majeure : le pacte embrasse l'ensemble du champ migratoire. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de réformer le régime européen de l'asile, mais de couvrir l'ensemble des instruments dont nous disposons ou d'en développer de nouveaux. Le pacte contient d'abord une refonte du régime européen de l'asile. Je distingue ici trois sujets. Premièrement, nous ne pouvons laisser les États membres dits « de première entrée » subir seuls les conséquences de la géographie ils gardent notre frontière extérieure pour le compte de tous les autres. Cette réalité implique une politique de solidarité que la France soutient. Nous en avons montré l'exemple avec des pays comme la Grèce ou l'Italie. Deuxièmement, la disparité actuelle des pratiques n'est pas viable, qu'il s'agisse des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, des délais d'instruction des demandes ou même des taux de protection par nationalité. Il nous faut harmoniser tout cela. Troisièmement, les États membres, et notamment ceux qui, comme la France, sont les principaux destinataires des flux secondaires, doivent avoir la garantie

ils alimentent pendant des années des flux secondaires à travers l'Europe. Ce dernier point renvoie au deuxième aspect majeur du pacte, à savoir la protection de la frontière extérieure. Pour répondre au terrorisme islamiste, qui a frappé notre pays en 2015, nous avons procédé au rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, comme le permet le code Schengen. Or, pour conserver l'esprit de Schengen, le Gouvernement juge essentiel le règlement dit « filtrage », qui fait partie du pacte et qui instaurera à la frontière extérieure des obligations de contrôle beaucoup plus strictes. Le contrôle rigoureux de la frontière extérieure nous semble en effet être l'une des conditions de la solidarité à l'égard des États « de première entrée Enfin, le pacte traite la dimension extérieure des migrations, composante essentielle d'une politique migratoire efficace. Là encore, nous avons bien progressé. Je rappelle, par exemple, que l'Union européenne, notamment sous l'impulsion de la France, a adopté en 2019 un règlement instituant, à l'échelon européen, un mécanisme dit «visa-réadmission» il s'agit de restreindre l'accès aux visas dans les pays qui ne coopèrent pas suffisamment avec nous en matière de réadmission. Vous le savez, c'est un sujet d'actualité. D'une manière générale, la France estime que l'Union européenne doit mener un dialogue plus exigeant et mutuellement bénéfique avec les pays d'origine et de transit. Le Conseil européen a adopté en juin dernier des orientations ambitieuses en ce domaine. Dans ce dialogue, nous croyons que toutes les questions doivent être abordées : la coopération en matière de réadmission, mais aussi la gestion concertée des flux migratoires, le soutien opérationnel et financier à ces pays, la lutte contre les trafics d'êtres humains et les réseaux de passeurs ou encore le développement économique. Nous sommes à quelques semaines seulement de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Les objectifs du Gouvernement sont de construire une Europe plus solidaire et plus souveraine. Le pacte sur les migrations et l'asile, dans un domaine important pour les Européens, y contribue. La France assurera avec détermination, pendant les six mois de sa présidence, la conduite des négociations européennes. Le pacte peut être une étape dans la construction d'un espace de libre circulation plus sûr et dans la mise en place de partenariats féconds avec les pays d'origine et de transit des migrations.

À quelques mois de l'élection présidentielle, la droite veut nous refaire le coup de Sarkozy en 2007 : montrer les muscles et parler fort contre l'immigration. Mais on connaît le truc : vous nous aviez promis le Kärcher

de clandestins- soit l'équivalent de la population du Danemark -entrés en Europe lors de la crise de 2014, déclenchée par votre grande amie Angela Merkel lorsqu'elle a laissé entrer de soi-disant réfugiés syriens, qui se sont révélés, pour certains, de vrais terroristes, le 13 novembre 2015, ou de vrais violeurs, le 31 décembre suivant, à Cologne.

de tous ceux qui agressent, tuent, violent ou font pire encore, à retirer la nationalité aux binationaux qui commettent un crime, à rétablir la double peine. Croyez-moi, tous nos problèmes financiers liés à l'insécurité seront alors en grande partie résolus. On aura bien un petit pic d'émissions de CO2 à cause des charters, mais, pour chaque personne expulsée, je m'engage à ce que nous replantions un arbre dans les banlieues, redevenues françaises. Nous avons déjà un haut-commissariat à la relance ; dans quelques mois, j'espère que nous aurons un haut-commissariat à la « remigration les répartir ; ils doivent repartir ! Madame la ministre, ne pensez-vous pas que le temps soit venu de tirer les enseignements de quarante ans de folle politique d'immigration. Loin d'être une richesse pour notre pays, l'immigration est en train de le ruiner ; ; loin d'être une chance, elle est un véritable fléau pour les Français. Le seul pacte que nous devons appliquer de toute urgence est celui du grand rapatriement des étrangers vers leur pays d'origine.

passent par l'instauration d'une solidarité forte entre les États membres de l'Union européenne. Enfin, les gesticulations nationales conduisent à des transferts de problèmes d'un voisin à un autre, aggravent la situation humanitaire, et portent atteinte à la libre circulation dans l'espace Schengen : elles ne sont donc pas la solution. Pourtant, madame la ministre, un ancien responsable européen, Michel Barnier, a évoqué un « bouclier constitutionnel » pour éviter finalement de respecter le droit européen sur ce sujet. D'autres gouvernements, actuellement, se livrent à des actions en violation flagrante du droit européen et des droits humains. Je pense en particulier à la Pologne, qui fait face à une attaque hybride d'un État passeur, mais qui n'en doit pas moins respecter le droit européen. Cette évolution est très préoccupante, madame la ministre. Ma question est simple : à quoi cela sert-il de négocier un nouveau pacte européen qui s'appuie sur des convergences fortes entre les États membres si, à l'avance, un nombre important d'États annoncent qu'ils ne le respecteront pas, et qu'il n'y a pas de clause claire obligeant chaque État à respecter les obligations qu'il prendra ?

prend précisément acte du fait que les règles existantes n'ont pas été efficaces. Je vous rejoins donc sur le constat que vous posez. Ce pacte propose justement de repartir sur de nouvelles bases par rapport au paquet Asile de 2016. 2016. Nous partageons avec nos voisins européens un espace de libre circulation. Cela implique de se doter de règles communes : les deux nous semblent étroitement liés. Cela implique aussi de définir des solutions ensemble, car nous appelons de nos voeux la construction d'une Europe qui puisse protéger avec des règles communes.

y compris celui du contrôle de la frontière extérieure. Nous continuerons à faire valoir les intérêts de la France et cette position dans cette négociation. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour la réplique. Madame la ministre, pensez-vous que, par exemple, les gesticulations auxquelles nous nous livrons à la frontière franco-espagnole pour repousser le problème en Espagne

Madame la ministre, la question migratoire fait aujourd'hui partie du quotidien de l'Union européenne. Plusieurs de ses États membres, dont la France, se situent en première ligne de ces flux, et payent le tribut d'une politique de migration et et d'asile européenne largement insuffisante au regard des enjeux qui restent devant nous. Afin de poursuivre et même d'accélérer les efforts mis en oeuvre depuis 2016, la Commission européenne a présenté voilà un an son pacte européen pour l'asile et les migrations, qui vise à proposer un système global de gestion des flux migratoires aux frontières de l'Union européenne, articulé autour de trois axes : le renforcement des frontières extérieures ; un partage plus équitable des responsabilités et de la solidarité ; le renforcement de la coopération avec les pays tiers. Ce pacte s'est révélé relativement ambitieux. Toutefois, son adoption est aujourd'hui au point mort. Les négociations n'ont pas été engagées et chacun semble préférer se renvoyer la balle, quitte à rester au faute d'accord. Le Parlement européen lui-même a accueilli froidement ce texte, notamment en raison du maintien du principe de responsabilité de l'État membre de première entrée, qui a montré toutes ses limites lors des vagues migratoires successives, laissant les pays concernés livrés à leur sort. Dans moins de trois mois, la France sera amenée à jouer un rôle moteur au sein de l'Union européenne, en assurant la présidence du Conseil de l'Union européenne. Dans ce cadre, madame la ministre, sera-t-elle en mesure de débloquer les négociations pour l'adoption du pacte européen pour l'asile et les migrations ? De quelle solution alternative disposons-nous si le blocage venait à perdurer ?

dont la négociation a déjà atteint un certain degré de maturité lors du premier cycle des trois premières années de négociation : sur les items du règlement Réinstallation et Eurodac, et sur les directives Accueil et Qualification. vous avez parfaitement raison de souligner que des points de blocage substantiels demeurent encore dans ces échanges. Ainsi, les États membres de première entrée, notamment Chypre, l'Espagne, la Grèce, l'Italie et Malte, demandent de la part de leurs partenaires davantage de garanties en matière de solidarité. Ils se montrent particulièrement réticents à mettre en place des procédures frontalières obligatoires sur leur sol. À l'inverse, des États comme la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, la Tchéquie, marquent leurs réserves sur le volet solidarité du pacte. Ils plaident pour une plus grande flexibilité, pour ne pas être contraints de procéder eux-mêmes à des relocalisations. Les États membres de destination que sont l'Allemagne, la Belgique, la Finlande, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Irlande et la Suède ont des positions nuancées et constructives dans la négociation. Comme eux, je le crois, les autorités françaises sont attachées aux quatre volets principaux du pacte que sont la solidarité,

Nous traversons, et nous allons traverser des tensions démographiques, géopolitiques, climatiques, qui entraîneront des mouvements de population plus importants que ce que nous connaissons actuellement. l'Union européenne doit être un espace de protection, de liberté et de stabilité. Nous devons avancer, évidemment, sur les mécanismes de coordination entre États lors des crises migratoires,

tant ces sujets relèvent de la souveraineté nationale, des gouvernements en place et de la situation politique du pays concerné. Il n'est que de voir ce qui s'est passé lors de la crise syrienne. Cependant, nous devons travailler à un cadre commun d'harmonisation du droit d'asile à l'échelle européenne. En ce qui concerne les frontières nationales, avec Schengen, nos frontières ne sont plus avec l'Allemagne et la Belgique, mais aux portes de l'Estonie, de la Grèce, ou à la pointe de l'Italie. Pour porter une vraie politique d'immigration, il faut s'en donner les moyens.

je vous remercie de votre question. Le renforcement de Frontex est largement entamé. Nous en avions d'ailleurs débattu ici. Depuis sa création en 2004, l'agence a vu ses moyens et ses compétences se renforcer considérablement, notamment avec le règlement européen du 14 septembre 2016, puis avec l'adoption du dernier règlement en date, le 13 novembre 2019. Ce dernier texte, relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, a pour objectif de maintenir la sécurité des frontières extérieures de l'Union européenne, mais aussi de permettre à Frontex de passer d'un rôle réactif à un rôle proactif, en prévoyant, par exemple, des déploiements à long terme, plutôt que de toujours réagir à des situations d'urgence. Il s'agit de renforcer la résilience des autorités nationales.

avec les directeurs exécutifs des neuf divisions de l'agence. Cette réorganisation s'accompagne d'une augmentation considérable des moyens humains. Le point central est la création d'un corps de garde-frontières et de garde-côtes européens de 10 000 agents, répartis en quatre catégories. Frontex

Les États membres de l'Union font en effet face à une crise migratoire larvée, dont le paroxysme a été atteint entre 2015 et 2016, avec, notamment, la crise syrienne et ses conséquences sur les arrivées incontrôlées sur le continent. Cette crise a agi comme un révélateur de nos impuissances. Une approche globale est donc indispensable pour surmonter nos divisions internes et être en mesure de proposer une réponse commune aux personnes qui affluent vers nos frontières extérieures. Ce défi est d'autant plus stratégique que l'Europe est encore l'une des premières destinations des flux migratoires dans le monde. Le 23 septembre dernier, la Commission a proposé une version revisitée et révisée de son pacte européen pour l'asile et les migrations. Cette version vise à surmonter les blocages ayant fait échouer les conclusions du paquet Asile présenté en 2016. Certes, ce pacte européen assume une approche globale, opportune et bienvenue. Il est en effet nécessaire d'apporter de la cohérence aux efforts déployés pour le contrôle aux frontières, la migration et l'asile, ainsi que de rétablir une confiance mutuelle, qui a tant fait défaut ces dernières années Je note donc un changement de ton et de perspectives. Il était temps, car l'irénisme et le déni de réalité qui ont accompagné le laisser-aller et le laisser-faire ayant dominé à Bruxelles sur ces questions ont fait beaucoup de mal. Les objectifs affichés du nouveau pacte, tels que la nécessité de renforcer les partenariats et la coopération des pays tiers, se veulent rassurants, mais ce n'est pas la première fois que l'objectif de renforcer les frontières extérieures est affiché. Ce nouveau paquet introduit par ailleurs un nouveau critère de la définition de l'État membre responsable d'une demande d'asile. Le principe de pays « de première entrée » n'est pas abrogé, mais il vient désormais en dernière position. La modification des

la nécessité de rechercher un équilibre entre les États membres. Ce principe guide les discussions qui ont eu lieu jusqu'à présent et guidera notamment l'engagement de la présidence française de l'Union européenne. C'est exactement pour faire face aux défis que vous avez mentionnés que la Commission européenne a proposé

européenne, ambitieuse et, surtout, efficace. C'est grâce à nos règles de responsabilité, qui seront contenues dans ce pacte, auquel, je l'espère, les États adhéreront, que la France devrait recevoir moins de demandes d'asile, mécaniquement. Surtout, elle devrait recevoir des

de peloton, à côté de l'Autriche et de la Pologne. Et nous ne voyons guère ce qui changera avec ce nouveau pacte, sinon la menace de faire porter une partie des coûts de la politique de non-accueil sur les pays européens récalcitrants au devoir d'asile et de solidarité. Ce pacte, en vérité, n'est pas cadré pour l'accueil, car, pour assumer cette exigence, nul besoin de nouveau pacte. La France pourrait, par exemple, activer la directive de 2001 sur la protection temporaire, qui permet déjà aux pays européens, en cas de situation d'urgence humanitaire ou d'afflux massif de réfugiés, de mettre en place un système de solidarité, d'accueil et de relocalisation des personnes. Madame la ministre, pourquoi la France n'a-t-elle jamais proposé l'activation de cette directive auprès de l'Europe, ni en février 2020, lorsque la Turquie, par chantage, expulsait des migrants syriens vers la Grèce, ni récemment, à Kaboul, lorsque des milliers d'Afghans étaient livrés aux talibans ? Plutôt que de refaire un pacte, qu'attendent l'Europe et la France pour activer les textes existants ? La parole

dans l'Union européenne, de ressortissants étrangers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine, notamment pour les raisons que vous avez évoquées : guerre, violences, violation des droits humains. Elle met en place une protection immédiate et temporaire pour ces personnes déplacées. Les bénéficiaires de la protection temporaire ont la possibilité de déposer une demande d'asile, et le pays de l'Union européenne qui a accueilli la personne est responsable de l'examen de la demande dans le temps. S'agissant particulièrement de la situation afghane, à ce stade, l'activation de cette protection temporaire immédiate n'est pas apparue nécessaire, parce que la France a évacué et accueilli plus de 2 600 personnes venant d'Afghanistan

Cette mobilisation se poursuit aujourd'hui pour permettre un enregistrement rapide de leur demande d'asile dès la fin de la quarantaine qu'ils doivent subir à leur arrivée pour raisons sanitaires. Je veux saluer le travail de la délégation interministérielle à l'accueil et à

À ce stade, donc, le régime de la protection temporaire n'a pas besoin d'être activé s'agissant des personnes venant d'Afghanistan. Nous réévaluerons sa nécessité en fonction de l'évolution de la situation sur place et des flux d'arrivées de personnes qu'elle engendre. La parole

Nous poursuivons tristement notre sous-traitance honteuse en confiant aux pays tiers, dont la Turquie, la gestion des personnes migrantes. Comment les États ont-ils fait front pour accueillir les Afghans ? En se livrant à des comptes d'apothicaires, en mobilisant des garde-frontières et en déléguant notre dignité aux pays voisins. Allons-nous laisser adopter des dispositions éparses et parmi les plus répressives d'un pacte qui ne répond en rien aux exigences humanitaires actuelles ? Pis, il propose un nouveau règlement relatif aux situations de crise et de force majeure, et prévoit des dérogations aux règles qui s'appliquent en matière d'asile, en suspendant, par exemple, l'enregistrement des demandes d'asile pour une durée d'un mois maximum. Cette mesure entérine des pratiques contraires au droit international et européen, auxquelles a recouru notamment la Grèce, début mars 2020, pour refouler les migrants venus de Turquie. Alors que ce nouveau pacte veut tirer les leçons du passé, il choisit, à l'approche de catastrophes humanitaires à venir, un mécanisme pour que l'Union se dérobe à ses responsabilités. Les crises que nous allons vivre ne peuvent s'accommoder de cette démission. Les réfugiés climatiques seront 250 millions en 2050, d'après l'ONU, sans parler des crises politiques qui rebattront régulièrement les cartes des équilibres régionaux et précipiteront dans l'exil nombre de familles. Madame la ministre, quelle sera la position de la France sur ce sujet ?

Le Danemark a adopté une législation très différente en matière de droit d'asile, en procédant à ce que les Danois appellent une externalisation. Quelle est l'opinion du Gouvernement français à cet égard ?

un projet de loi qui vise à externaliser sa politique d'asile dans des États tiers, avec quelques exceptions dans ce dispositif, notamment pour les personnes gravement malades, les demandeurs dont la famille réside légalement au Danemark et les mineurs non accompagnés dont les parents seraient établis en Europe. À ce stade, très sincèrement, il reste difficile de procéder à une analyse juridique définitive de la loi danoise, puisqu'elle se limite à prévoir la possibilité de transférer les demandeurs d'asile dans un État tiers, et que la loi danoise ne précise pas les modalités de cette mise en oeuvre. Au regard du droit européen, le Danemark est membre de l'espace Schengen, mais il ne participe pas, en raison de son option de retrait de toutes les mesures de justice et d'affaires intérieures, au régime d'asile européen commun. Il applique uniquement les règlements dits Dublin III et Eurodac, et conserve donc, en droit,, la possibilité d'établir son propre accord de réadmission avec des pays tiers. Toutefois, je précise que la loi danoise ne pourrait respecter les engagements européens et internationaux du Danemark qu'à condition que les accords conclus avec les pays tiers concernés comportent des garanties solides, notamment sur le plan du respect des droits fondamentaux des personnes. La parole

notamment l'Allemagne, ce qui entraîne des mécanismes dits de rebond. Cela fait partie des solutions qui permettraient d'améliorer la situation, sachant que, très probablement, l'atténuation des effets de la pandémie et le retour des déplacements conduiront notre pays à connaître une situation tendue sur ces sujets dans les mois à venir.

un défi qui appelle un approfondissement de sa politique commune en la matière, notamment au regard des crises géopolitiques qui ouvrent régulièrement de nouvelles voies de migration, ou encore de l'instrumentalisation sans complexe des migrants par certains pays, comme récemment la Biélorussie. Aussi mon groupe est-il ouvert aux propositions du pacte européen pour l'asile et les migrations, tout en étant inquiet des positions de certains États membres, qui risquent de retarder l'adoption des outils dont l'Europe a pourtant besoin très rapidement. En attendant, je souhaiterais évoquer moi aussi les moyens d'un instrument existant, Frontex, dont le travail est à la fois reconnu et critiqué. Je pense notamment aux observations de la Cour des comptes, ainsi qu'aux accusations de violation des droits de l'homme visant l'agence. Son règlement fondateur a été modifié à quatre reprises, en 2007, 2011, 2016 et 2019. Il pourrait l'être une nouvelle fois par le futur pacte. Au fil de la pression migratoire, les missions de Frontex ont été ainsi enrichies. Les agents sont aujourd'hui compétents pour enregistrer et identifier les migrants, ainsi que pour coordonner les opérations de retour. Dans ces conditions, madame la ministre, les moyens de Frontex sont-ils suffisants en capacité opérationnelle ? Les personnels sont-ils formés pour leurs nouvelles missions ? La parole

précédemment, je veux rappeler que le renforcement de Frontex est en cours, notamment avec l'adoption du dernier règlement, en date du 13 novembre 2019, qui permet à Frontex de passer d'un rôle réactif à un rôle proactif, et qui s'accompagne d'une véritable augmentation de ses moyens humains. Nous en avions d'ailleurs débattu ici même, me semble-t-il, voilà quelques semaines ou quelques mois. Le point central est la création d'un corps de garde-frontières et de garde-côtes européen,

2027. Bien sûr, cette montée en puissance doit s'accompagner de la formation adéquate des personnels. Je veux vous rassurer, monsieur le sénateur, la France veille et va veiller à ce que ce soit bien le cas, et des évaluations seront conduites année après année. La parole

de celle qui ressort des propos outranciers à visée électorale tenus par certains. Nous sommes bien loin d'une supposée immigration massive. Il n'en reste pas moins que, pour les principaux intéressés, ceux qui fuient la guerre et les persécutions, obtenir l'asile est un véritable chemin de croix. Face à la crise migratoire, les États membres n'ont pas su, ou n'ont pas voulu faire preuve de solidarité. Les dispositions législatives et réglementaires européennes ont montré leurs limites et la Commission, pour dépasser les difficultés, a lancé l'élaboration d'un nouveau pacte. Aujourd'hui, la situation est bloquée, et ce sont des logiques nationales qui s'affrontent et se substituent à l'approche européenne commune. Trois groupes se distinguent : les pays du Groupe de Visegrád, qui s'opposent aux règles de solidarité ; les pays « de première entrée », qui considèrent à juste titre que le nouveau pacte n'allégerait pas la pression qu'ils subissent ; et un groupe intermédiaire de pays, dont la France, qui cherchent un compromis. Madame la ministre, le pacte européen pour l'asile et les migrations est dans l'impasse. Par ailleurs, il contient un certain nombre de sujets qui ne peuvent pas être acceptés,

Ce pacte fait l'impasse sur la solidarité, aucune obligation ne reposant sur les États membres pour relocaliser les personnes d'un pays vers un autre, mais instaure des parrainages au retour, exonérant les États de leurs obligations. l'asile et les migrations pourrait être adopté, abandonné ou scindé par thèmes pour pouvoir faire avancer les sujets plus consensuels, comme la création de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile ? Ne pensez-vous pas qu'il serait préférable de changer d'orientation et de privilégier une coopération renforcée avec les États membres volontaires et solidaires, en utilisant par ailleurs le bâton de la conditionnalité des aides pour ceux qui ne jouent pas collectif ?

Nous sommes en train de bâtir un autre programme pour la présidence française de l'Union européenne, et ce en concertation étroite avec nos partenaires, à commencer par la présidence slovène, la Commission européenne et le secrétariat général du Conseil.

Vous testez d'ailleurs, à quelques mois de l'élection présidentielle, la pression sur les pays d'origine par la politique des visas. Cependant, qu'en est-il pour ceux qui sont sur le territoire européen ou qui réussiront à y entrer pour tenter de rejoindre le Royaume-Uni ? Je pense à la situation dans la zone Manche-mer du Nord, dont le département du Calvados fait partie : une hausse significative des traversées y est constatée depuis plusieurs semaines. Certaines communes, de la côte normande aux rivages du Pas-de-Calais, sont en première ligne et récoltent les désagréments d'un contexte qui dure de fait depuis plusieurs années. Depuis le Brexit, les autorités britanniques ont durci le ton en matière migratoire. Elles viennent en outre d'approuver une nouvelle stratégie de refoulement des embarcations de migrants vers la France. Dès lors, madame la ministre, face à un Royaume-Uni qui

Nous aurons alors à engager des négociations avec le Parlement européen, mais aussi à faire progresser le règlement dit filtrage, qui instaure des procédures plus rigoureuses à la frontière extérieure. Enfin, en dehors du pacte, il nous reviendra de diriger la négociation sur le règlement Schengen à venir, appelé à réformer le régime des contrôles aux frontières extérieures. La parole

Jean-Michel Arnaud. Madame la ministre, en dépit du règlement dit Dublin III, une partie significative des demandes d'asile ne sont pas traitées par les États d'entrée, à la fois par manque de volonté politique et par manque de solidarité européenne. Cela a notamment pour effet un accroissement des mouvements secondaires de migrants entre les États au sein de l'Union européenne. En France, dans mon département des Hautes-Alpes, par exemple, ce problème est particulièrement aigu. En 2020, plus de 11 000 passages illégaux ont été répertoriés entre l'Italie et la vallée de Briançon. Ces passages, qui s'effectuent principalement par le col de l'Échelle, devenu tristement célèbre, ont pour destination finale Londres, Calais. La pression migratoire locale est accentuée par l'inadéquation des moyens alloués à la police aux frontières, ce qui ne permet pas toujours d'assurer un accueil digne, à la hauteur de nos idéaux humanistes. vous l'avez compris, la dérégulation du système migratoire ne peut plus durer. Les facteurs de difficulté résident notamment dans le traitement des demandes et dans l'exécution des obligations de quitter le territoire français Le pacte européen pour l'asile et les migrations esquisse quelques avancées qu'il convient de concrétiser. Mes questions sont donc les suivantes. Alors que les obligations de quitter le territoire français sont souvent difficiles à exécuter, quel sera l'apport du coordinateur de l'Union européenne chargé des retours ?

Monsieur le sénateur Arnaud, la stratégie de l'Union européenne en matière de retour volontaire et de réintégration est un objectif clef du pacte européen pour l'asile et les migrations. Elle définit notamment les mesures pratiques pour pouvoir consolider le cadre juridique et opérationnel des retours volontaires depuis l'Union européenne. Cependant, les écarts entre les procédures d'asile et de retour, la difficulté d'empêcher la fuite des personnes, les capacités administratives limitées pour assurer le suivi des décisions de retour, expliquent notamment le faible succès des programmes d'aide au retour volontaire jusqu'à présent. Grâce à son mandat élargi, l'agence Frontex est en mesure d'aider les États membres à tous les stades du processus de retour volontaire et de réintégration. européenne chargé des retours et le réseau de haut niveau pour les retours pourront apporter un soutien technique supplémentaire aux États membres pour regrouper les différents stades de la politique de l'Union européenne en matière de retour.

S'agit-il au contraire des visas de court séjour Schengen ? Dans ce cas, ce serait peu opérant, puisqu'il suffirait que les demandeurs de visas s'adressent à d'autres pays européens.

Ces mesures sont justifiées par le niveau très insatisfaisant de la coopération avec les pays du Maghreb, et ce depuis plusieurs mois : seulement 105 Marocains ont été éloignés entre le 1 janvier et le 31 août 2021, contre 908 en 2019

Cette situation est d'autant plus incompréhensible pour nos concitoyens que la pression migratoire en provenance de ces trois pays reste élevée et que ces flux peuvent concerner des personnes impliquées dans des troubles à l'ordre public. Ces mesures sont d'application immédiate. Elles sont réversibles dans le temps : si nos partenaires font de réels efforts pour améliorer leur coopération, nous suspendrons l'application de ces mesures. Des efforts ont d'ailleurs déjà été constatés en Tunisie,

je vous le dis : la France visera en priorité les milieux dirigeants, qui sont les premiers responsables de cette situation de blocage. La parole

Lavarde. Madame la ministre, voilà six ans, face à une crise migratoire sans précédent, les citoyens européens découvraient avec effarement l'impréparation des États membres, totalement dépassés par l'ampleur des flux. à enregistrer les arrivants ou leur refus de le faire ont largement contribué au chaos. Le faible niveau d'équipement de certains États, la fragmentation des différentes bases de données numériques et leur utilisation inégale ont été sources de difficultés dans la gestion de la crise. Ces difficultés n'étaient pas nouvelles : elles avaient déjà été identifiées dans un rapport de 2007, qui avait accompagné la modification du règlement Eurodac intervenue en 2008. La création de nouveaux systèmes d'information et leur mise en interopérabilité ont donc été logiquement des chantiers prioritaires ces dernières années.

les contrôles aux frontières extérieures et la gestion de l'immigration. Elle consistera à faire dialoguer différents systèmes d'information européens, notamment les systèmes d'information Schengen et Eurodac. Elle permettra aux autorités de contrôle aux frontières, d'immigration et de sécurité intérieure d'obtenir en une seule requête des informations détaillées provenant de tous les systèmes d'information pertinents auxquels elles ont accès. L'identification des ressortissants de pays tiers sera d'ailleurs facilitée grâce à la possibilité de comparer les données biométriques provenant de différents systèmes d'information. Les autorités pourront par exemple détecter les cas d'identités multiples ou de fraude à l'identité. L'interopérabilité, qui devra être mise en oeuvre à la fin de l'année 2023, après la mise en oeuvre des nouveaux systèmes d'information aux frontières et la révision des systèmes existants, apportera donc une plus-value majeure aux contrôles aux frontières et à la sécurité des citoyens européens. La parole

dans le cadre du pacte européen pour l'asile et les migrations, la Commission européenne propose de bâtir un nouveau système commun de gouvernance. Celui-ci s'appuierait sur l'élaboration de stratégies nationales et européennes, ainsi que sur de nouveaux mécanismes de suivi et d'évaluation des politiques nationales. Au vu des dysfonctionnements profonds observés depuis longtemps dans certains États membres en ce qui concerne la maîtrise des frontières extérieures et la gestion des flux migratoires, ce contrôle accru et cette coopération renforcée étaient devenus indispensables. Cela paraît toutefois encore insuffisant. Gardons en effet à l'esprit que l'espace Schengen n'est pas seulement un espace de liberté, c'est également et surtout un espace de souveraineté en commun. En conséquence, il ne devrait rassembler que les seuls États capables d'assumer cette souveraineté en gérant efficacement leurs frontières, même si la solidarité européenne doit naturellement s'exprimer en cas de crise exceptionnelle. Ainsi, les États membres qui ne seraient pas en mesure de respecter leurs obligations ou qui ne donneraient pas suite aux recommandations formulées pour pallier leurs défaillances devraient-ils pouvoir être sanctionnés, voire, en dernier recours, suspendus de l'espace Schengen. Aucune procédure de ce type n'est toutefois évoquée à ce jour, que ce soit dans le pacte ou dans la stratégie présentée au mois de juin dernier par la Commission européenne pour le renforcement de l'espace Schengen. Le Président de la République affirmait, avant les dernières élections européennes, sa volonté de « remettre à plat » l'espace Schengen et insistait sur le fait que « tous ceux qui veulent y participer doivent remplir des obligations de responsabilité Madame la ministre, ma question est simple : la France plaidera-t-elle pour la mise en place d'un régime de sanctions spécifiques à l'encontre des États qui ne se donneraient pas les moyens de contrôler efficacement les flux migratoires ?

Cela nécessite une confiance mutuelle qui doit s'appuyer sur un certain nombre d'éléments objectifs et de décisions. C'est pourquoi la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen dans le domaine des frontières extérieures fait l'objet d'une évaluation régulière de chaque État membre. Les recommandations des rapports d'évaluation doivent d'ailleurs donner lieu à un plan d'action de l'État concerné pour y remédier. En cas de défaillance grave, qui mettrait en péril le fonctionnement de l'espace Schengen, la Commission européenne peut recommander à l'État membre évalué le déploiement d'équipes européennes de garde-frontières sous l'égide de l'agence Frontex. Le Conseil peut aussi en dernier recours, pour protéger les intérêts communs au sein de l'espace Schengen, recommander à des États membres de réintroduire le contrôle à leurs frontières intérieures. processus, un État persistait à ne pas remédier à une défaillance qui aurait été constatée, la Commission européenne pourrait introduire contre lui une procédure d'infraction devant la Cour de justice de l'Union européenne. Ainsi, il n'est pas possible que des défaillances graves du contrôle aux frontières par un État demeurent inconnues de ses partenaires et ne donnent pas lieu à une réaction. Monsieur le sénateur, j'espère avoir répondu à votre question. La parole

quelle politique vous voulez réellement en matière migratoire et en matière de droit d'asile, sans vous cacher sous la couverture européenne, qui, malheureusement ou heureusement, est assez peu efficace en ce moment ?

par le ministre de l'intérieur de l'époque, Gérard Collomb, et a défini les grandes orientations du Gouvernement. Celles-ci étaient conformes à la ligne directrice du Président de la République, qui a prôné un équilibre entre humanité et fermeté. L'humanité, c'est le respect des droits humains, le respect des droits de chacun, le respect de la Convention de Genève

D'autres font en revanche l'unanimité, telles que la nécessité de renforcer la dimension extérieure de la politique migratoire européenne. Bien évidemment, la recherche d'un accord sur l'ensemble ne doit pas être abandonnée, mais l'accent doit être mis sur ces propositions consensuelles pour obtenir,, un renforcement de notre politique migratoire en cas d'échec des négociations. la décision de la France de durcir la politique des visas à l'égard des pays du Maghreb ne peut qu'être bienvenue. Il est toutefois regrettable qu'elle intervienne si tard, alors que cela fait de nombreuses années que les pays du Maghreb rechignent à délivrer des laissez-passer consulaires. Je comprends bien que l'utilisation des voies diplomatiques devait primer dans un premier temps, mais ce phénomène n'est pas nouveau et aurait pu être réglé bien plus tôt. Certes, mieux vaut tard que jamais

Il est désormais nécessaire que l'Union européenne durcisse le ton face aux pays peu coopératifs. Une décision unilatérale de la France ne suffira pas à elle seule à remédier aux lacunes que l'on constate.

L'utilisation de l'ensemble des leviers dont nous disposons est donc essentielle. Il faut rechercher une synergie et se coordonner avec les autres États membres en s'appuyant sur les relations privilégiées que chacun entretient avec certains pays pour mieux négocier les accords d'association. Je pense également à la conditionnalité des aides au développement à des accords de coopération en matière d'accueil, de retour et de réinstallation. Une meilleure quantification et un meilleur suivi de la coopération des États tiers permettraient aussi de moduler les aides et les quotas de visas en fonction de leurs efforts. Aussi, madame la ministre, la France se positionnera-t-elle en faveur d'un durcissement de la politique européenne envers les pays peu coopératifs, tout en renforçant la dimension extérieure de la politique migratoire, dans le cadre de sa présidence du Conseil européen et dans les négociations sur le pacte européen pour l'asile

nous privilégions avant tout le dialogue avec les pays en question, conscients que nous sommes des contraintes qui peuvent peser sur leur action et de la complexité de leur situation intérieure. Néanmoins, quand la non-coopération s'installe dans la durée, ce que nous avons étayé avec des chiffres, elle n'est plus justifiée et il nous faut alors prendre des mesures claires et assumées, comme nous l'avons fait récemment à l'encontre du Maghreb. À l'échelle européenne, nous soutenons la mise en oeuvre de partenariats équilibrés qui soient mutuellement bénéfiques entre les pays d'origine et de transit pour répondre aux pays coopératifs par une offre ouverte en matière d'aide au développement, de relations commerciales, de renforcement capacitaire et de voies légales de migration. Au contraire, nous devons conduire un dialogue exigeant avec les pays qui ne le sont pas et mobiliser tous les instruments dissuasifs possibles- visas, mobilités, etc. C'est dans cet esprit que nous aborderons la présidence du Conseil de l'Union européenne. En conclusion